En application de l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, M. le président du Sénat a reçu de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, une communication de laquelle il résulte que, à la suite des opérations électorales du dimanche 17 décembre 2017, M. Yves Bouloux a été proclamé sénateur de la Vienne, Mme Évelyne Perrot a été proclamée sénatrice de l'Aube et Mme Dominique Verien, sénatrice de l'Yonne. Le mandat de nos collègues a débuté ce lundi 18 décembre à zéro heure. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur le second projet de loi de finances rectificative pour 2017 n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ne nous y trompons pas : c'est un vrai texte de décentralisation que nous examinons, après l'accord survenu

L'ordonnance que nous devons ratifier aujourd'hui doit entrer en vigueur le 1janvier 2018. Son contenu a été amélioré

de participer à des sociétés publiques locales dans le cadre de sa mission de promotion du site de la Défense et pour lui donner des moyens d'attirer de nouvelles entreprises et de nouveaux investisseurs. C'est

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, mesdames, messieurs les sénateurs, nous revenons devant la Haute Assemblée

ensemble pour parvenir à cette solution consensuelle. À la suite d'une ordonnance signée le 3 mai 2017 par le précédent gouvernement, quelques jours avant l'élection présidentielle, nous avons repris ce dossier qui avait été déjà très largement engagé sous le quinquennat précédent. Comme vient de le relever à juste titre le président de la commission des lois, il s'agit d'une d'une opération de simplification et de regroupement de deux entités, l'EPADESA et DEFACTO, pour donner plus d'efficacité

de permettre aux collectivités locales d'assurer la responsabilité pleine et entière de la gestion et du développement de ce quartier d'affaires. Bien

de surveillance à l'intérieur du périmètre et aussi de développement. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement, par ma voix, indique son accord sur les conclusions de la commission mixte paritaire en invitant

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, saluons ensemble la qualité du travail parlementaire qui a été ici réalisé, dans la clarification des périmètres d'intervention du nouvel établissement public Paris La Défense, dans la prise en compte des difficultés liées à l'insuffisance des investissements au cours des dernières années et dans le tracé des lignes de démarcation mettant au clair les responsabilités de l'État aménageur et des collectivités territoriales gestionnaires. Quand on veut se mettre d'accord, on peut ! Aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, tous ont reconnu la nécessité de regrouper dans une structure décentralisée les deux établissements chargés de l'aménagement et de la gestion de La Défense, afin de constituer un pilotage unifié du quartier d'affaires propre à pérenniser son activité et son attractivité. Ce postulat a fondé la nécessité d'une coopération territoriale approfondie, laissant une latitude appréciable aux collectivités concernées pour assurer, demain, les modalités pratiques de gouvernance du nouvel établissement. Leur capacité à moderniser et à sécuriser le quartier historique, à rénover ses accès et à l'ouvrir sur les territoires environnants constituera leur combat prioritaire. Nous apprécierons les résultats du nouveau dispositif essentiellement à la lumière de la réussite de cette mission, d'autant que, cette fois, une stratégie de développement pluriannuel a été élaborée. C'est un plan d'investissement, financé à hauteur de 360 millions d'euros au moins, sur dix ans, par les collectivités territoriales qui viendra désormais épauler la gestion coopérative de ce territoire d'intérêt national. À cet égard, la volonté du législateur est doublement satisfaite : par l'intégration de nouveaux instruments nécessaires au développement de cette place financière, mais aussi par le respect du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales dans l'esprit de la décentralisation. Nous ne pouvons pas sans cesse réclamer davantage de décentralisation et la contester lorsqu'elle advient. Quant aux dispositions qui pouvaient potentiellement créer des points de blocage-je pense notamment à la définition des périmètres d'intervention, modifiables par décret, ou à la possibilité de créer des filiales et d'acquérir des participations dans des sociétés publiques locales -, elles ont fait l'objet d'un accord entre nos deux assemblées. En définitive, c'est un texte de consensus, ce consensus qui a pu être dégagé en commission mixte paritaire, notamment grâce à l'esprit constructif de notre rapporteur, Mathieu Darnaud, que nous ne manquons pas féliciter pour l'important travail qu'il a abattu. C'est cet esprit qui est à l'origine de la modification de l'article 3 du projet de loi, afin de donner la possibilité à l'établissement public Paris La Défense, dans un cadre bien défini et sous certaines conditions, de recourir à des filiales pour engager une politique d'attractivité sur ce territoire.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons a pour objet de ratifier une ordonnance prise par le Président de la République François Hollande le 3 mai 2017. mai 2017. Déposé le 10 mai 2017 sur le bureau du Sénat, soit quatre jours avant la fin de la mandature présidentielle, il a pour conséquence de décentraliser totalement la gestion du quartier d'affaires de La Défense et procède à la fusion de l'établissement chargé de la gestion de son coeur historique et de l'établissement chargé de son aménagement et de celui d'une zone plus vaste, composée notamment du site d'opérations d'intérêt national Seine-Arche, couvrant un tiers du territoire de la commune de Nanterre.

L'objectif du Gouvernement, tel qu'il l'avait exposé au mois de mai 2016, était de confier la responsabilité principale de son pilotage et de son financement aux collectivités locales. Reprenant les conclusions d'un rapport rendu par les préfets de l'Île-de-France et des Hauts-de-Seine, ce texte avait pour ambition de « réinventer le modèle de la Défense pour rassembler tous les acteurs ». le texte soumis à notre approbation s'éloigne considérablement de cette première intention. En effet, le conseil départemental des Hauts-de-Seine disposera seul de la majorité des sièges du conseil d'administration du nouvel établissement public.

Cette gouvernance confiée exclusivement au conseil départemental des Hauts-de-Seine pose plusieurs problèmes, d'ordre juridique, politique et économique.

En droit, dans la rédaction actuelle du texte, tout se passe comme si la commune de Nanterre était subordonnée à une autre collectivité territoriale sur son propre territoire. Autrement dit, l'État a transféré ses prérogatives régaliennes à une seule collectivité, aux dépens d'une autre. Cette exclusivité nous semble discutable. À tout le moins, il eût été de bonne politique d'encadrer la relation de ces deux collectivités par des règles juridiques claires. Sur un autre plan, à l'échelle régionale et nationale, le quartier d'affaires de La Défense, au quatrième rang mondial par son importance, est considéré comme le « fer de lance de l'attractivité de la région-capitale La sortie probable du Royaume-Uni de l'Union européenne confère au quartier d'affaires une importance supplémentaire et impose de s'interroger sur sa capacité à accueillir de nouvelles activités. Cette réflexion est l'un des volets qui animent un débat plus général sur l'organisation de la métropole urbaine parisienne, sa gouvernance et son développement économique. Le Président de la République devrait annoncer prochainement ses propositions sur ce dossier. Il est donc surprenant que, sans attendre la clôture de ce débat, le présent texte ait fait le choix de confier au seul département des Hauts-de-Seine la gestion d'un quartier d'affaires dont tout le monde convient qu'il joue un rôle décisif dans le fait métropolitain. Par ailleurs, on peut se demander,, ce qu'il adviendrait de ce texte dans le cas d'une disparition des départements de la petite couronne ou de la fusion des Hauts-de-Seine et des Yvelines, sur laquelle le Gouvernement aura très prochainement à donner un avis. De façon plus générale, un examen comparatif des situations mondiales montre que les solutions adoptées pour la gestion des grands quartiers d'affaires reposent plutôt sur la coopération des collectivités principalement engagées dans la gestion du fait métropolitain.

On peut légitimement se demander si le département est le bon échelon pour assumer toutes les obligations qu'impose une telle responsabilité. Nous ne comprenons pas l'empressement à sceller le destin de ce quartier d'affaires, alors qu'un débat est en cours. Il est parfois urgent

conçoit le Centre national des industries et des techniques, dont la vocation reste encore hypothétique, mais dont l'acronyme, CNIT, restera lors de l'inauguration par le général de Gaulle, au mois de septembre 1958.

que vous pouvez toujours voir depuis la place de l'Étoile, dans cette belle et grande perspective. Aujourd'hui, soixante ans après, après, La Défense est le quatrième quartier d'affaires mondial et le premier quartier d'affaires européen, avec un bassin d'emploi de un million et demi de personnes.

l'État aménageur n'a pas fait son devoir. Les infrastructures en attestent : les quatorze tunnels qui passent sous le site ne sont pas aux normes de la directive européenne de 2004, la dalle est très fragilisée, le sous-sol est une friche non aménagée, comportant des espaces abandonnés et squattés, les conduites de fluides ne sont pas toutes identifiées, la desserte automobile est un labyrinthe inorganisé et instable, l'accès en sous-sol des tours est parfois décourageant. Je vous conseille de prévoir plusieurs jours pour retrouver un bureau à La Défense, tant l'accès est compliqué

de mon collègue Pierre Ouzoulias s'agissant de Nanterre. Je suis convaincu que les collectivités territoriales concernées sauront s'entendre, elles sont au sein de la même intercommunalité. Au demeurant, quand il a fallu construire la U ARENA

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui amenés à nous prononcer sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense. Nous parlons ici du premier centre d'affaires européen, La Défense représentant en effet 150 000 emplois et 3,2 millions de mètres carrés de bureaux. À l'aube du Brexit,

Cette réforme doit lui permettre à la fois d'être innovante et de consolider son rang de premier centre d'affaires européen. Soyons clairs, l'enjeu du premier centre d'affaires européen n'est pas seulement départemental : il est métropolitain, régional, national que nous ne pouvons pas sacrifier sur l'autel de l'efficacité toute notion de démocratie et de concertation. Pour garantir la mise en oeuvre d'une réforme ambitieuse, nous devons ainsi prendre le temps de la réflexion et associer tous les acteurs concernés, au premier rang desquels les communes.

Nous exprimons plusieurs désaccords avec le texte qui nous est aujourd'hui soumis. Nous avions d'ailleurs déposé deux amendements lors de la réunion de la commission mixte paritaire, mais, bien sûr, ils ont été rejetés. Le premier point de désaccord porte sur l'article 4, relatif à la composition du conseil d'administration. Il nous semble en effet primordial que le pluralisme

Le second point de désaccord est encore plus important et porte sur l'article 2, qui donne à l'établissement public Paris La Défense la possibilité d'intervenir en dehors de son périmètre historique d'intervention. Contrairement à ce qu'avait annoncé le précédent gouvernement dans un communiqué de presse du 27 mai 2016, l'établissement public n'aura pas l'obligation de passer des conventions d'aménagement avec les communes concernées. Je cite le communiqué : « Au-delà de ce périmètre, l'établissement disposera d'une compétence non exclusive d'aménagement et de gestion, définie par voie de conventions, notamment afin de garantir la poursuite par le nouvel établissement des opérations déjà engagées par l'EPADESA Or le texte que nous sommes appelés à voter prévoit le contraire. Il n'impose pas d'obligation de conventionner entre l'établissement public Paris La Défense et les communes, mais prévoit simplement un avis consultatif des acteurs concernés, et on connaît le sort de ces avis Je tiens à rappeler que le périmètre non exclusif de la gouvernance de l'établissement Paris La Défense concerne un tiers du territoire de la ville de Nanterre. Dès lors, pourquoi ne pas revenir à l'ambition initiale, à savoir une obligation de convention entre l'établissement public et la commune ?

Nous demandons simplement que la ville ait son mot à dire sur son territoire. Notre collègue Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques, l'a d'ailleurs parfaitement rappelé sur Public Sénat Public Sénat : « Au Sénat, nous considérons que les communes restent la cellule de base de la démocratie. » Dès lors, comment accepter qu'un établissement public puisse contrôler un tiers d'une commune sans même être obligé de passer des conventions avec elle ? chers collègues, le Président de la République avait annoncé lors de la campagne présidentielle une réforme territoriale d'envergure. Il avait indiqué : « Nous supprimerons au moins un quart des départements, là où ils peuvent être rapprochés de l'une de nos grandes métropoles. [ En concertation avec les élus, nous simplifierons l'administration territoriale en confiant aux services des métropoles les compétences des conseils départementaux où elles se situent. » Or nous

nous allons voter un texte dans la précipitation- à cet égard, je rappelle que la Cour des comptes a estimé que la décentralisation du quartier se faisait de manière trop rapide

Après la naissance de la métropole du Grand Paris, quel sera l'avenir de nos départements ? Quelle sera la gouvernance de l'établissement public Paris La Défense ? Ne devrions-nous pas attendre afin d'avoir une vision à long terme ?

Allons-nous barrer la route au juge administratif suprême ? Allons-nous le priver de ses fonctions consultative et juridictionnelle, au prétexte d'aller vite ? Mes chers collègues, la création d'un établissement public de cette envergure ne peut se faire dans la précipitation et sans réelle concertation.

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, l'article 55 de la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain a habilité le Gouvernement à créer, par ordonnance, par ordonnance, un établissement public unique se substituant aux deux établissements préexistants, DEFACTO et l'EPADESA, compétent à la fois pour l'aménagement, la gestion et la promotion du quartier d'affaires de La Défense. aménagement et gestion du patrimoine étaient répartis au sein de deux entités distinctes, ce qui, semble-t-il, n'a pas toujours été facile à gérer. Nous saluons l'unification de ces compétences entre les mains d'un seul acteur, car elle devrait favoriser la cohérence des actions menées. Ce pilotage unifié et un financement plus solide du quartier d'affaires ont été pensés à l'origine en vue de « pérenniser son attractivité ». Dans le contexte du Brexit et de la compétition européenne pour attirer les entreprises et les talents,

Cette vision n'est réalisable que si l'ensemble des acteurs concernés se mobilisent en faveur de la réussite de cet établissement, dans un contexte, je l'ai dit, très concurrentiel. Nous saluons ainsi la place plus importante accordée par ce texte aux collectivités, même si cela est contesté par certains, et la liberté accrue des acteurs locaux. En effet, l'administration du futur établissement sera assurée par un conseil d'administration de dix-sept membres, dont quinze représenteront les collectivités territoriales et leurs groupements : le département des Hauts-de-Seine, certes en tête, les communes de Courbevoie, de Nanterre et de Puteaux, la ville de Paris, le conseil régional d'Île-de-France et la métropole du Grand Paris, soit une véritable diversité, ce qui n'était pas le cas dans le montage précédent. Nous espérons que cette représentation accrue des collectivités s'accompagnera également d'une meilleure coordination avec l'État, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé, loin de là. Il faut mettre un terme à des désaccords qui ont pu être sources de fragilité et de lenteur, notamment en termes d'entretien et de gestion du site, afin que la nouvelle gouvernance soit l'ébauche d'une véritable « équipe de France », soudée autour de la promotion de l'excellence à la française. Les questions soulevées par ce texte portaient surtout sur le périmètre d'intervention du futur établissement et sur le rôle conservé par l'État. Sur le premier sujet, les périmètres ont été simplifiés et mieux définis par l'action conjointe

distincts, l'un exclusif en matière d'aménagement et de gestion portant sur le quartier historique de La Défense, l'autre partagé pour l'aménagement du territoire Seine-Arche. Des compétences nécessaires à la bonne gestion ont ont également été accordées au nouvel établissement, comme la vidéoprotection et, sous réserve de l'accord des maires concernés- ils restent bien dans la boucle -, des pouvoirs de police en matière de propreté de la voirie et de gestion des déchets. Nous saluons également le consensus qui a pu être trouvé sur la possibilité ouverte au futur établissement public de procéder, sous certaines conditions, à la création de filiales. En ce qui concerne le rôle joué par l'État, les débats sur les pouvoirs du préfet de région ont parfois illustré le malaise qui demeure souvent, dans dans notre pays, pas seulement à La Défense, en matière de coordination entre les différents acteurs concernés. Pour notre part, nous estimons que l'État a toute sa place dans la gouvernance du futur établissement public, compte tenu de son rôle, qui est certes local, qui est certes local, mais également régional et, évidemment, national. L'État doit pouvoir s'opposer aux décisions qui porteraient manifestement atteinte aux intérêts nationaux, en particulier à ses intérêts patrimoniaux, ou au bon fonctionnement des services publics. Néanmoins, nous pensons que la nouvelle rédaction de ce texte est plus équilibrée dans ce domaine

transmise au Sénat de la République le 10 mai. Si ce n'est pas de l'accélération de dernière minute, qu'est-ce que c'est ? J'ajoute qu'il est clairement indiqué est clairement indiqué dans l'ordonnance, telle qu'elle a été écrite le 3 mai : « Paris La Défense est administré par un conseil d'administration composé majoritairement de représentants du département des Hauts-de-Seine. En outre, sont représentées les communes de Courbevoie, Nanterre, Paris et Puteaux, ainsi que la région d'Île-de-France et la métropole du Grand Paris. » Il n'appartient pas au législateur de préciser le nombre

les mêmes choses. La discussion générale est close. Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte,

La séance est suspendue.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, après engagement de la procédure accélérée, mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement

cet accord indispensable pour protéger notre climat, ou plutôt, car l'expression est un peu faible, pour essayer de protéger tout ce qui est essentiel à nos yeux.

Certains avaient légitimement émis des doutes, pensant que ce projet de loi nous privait de marges de manoeuvre et que nous étions isolés dans notre démarche.

vers la sortie des énergies fossiles. Lors du même sommet, auquel je remercie certains d'entre vous d'avoir participé, nous avons aussi lancé la coalition vers la neutralité carbone. regroupe seize pays et trente-deux villes, qui s'engagent à publier le plus rapidement possible, étape après étape, une trajectoire vers la neutralité carbone à l'horizon de la moitié du XXI siècle. Ces pays, ces villes,

soit au pire neutre, au mieux négatif. Très concrètement, cela signifie que ces territoires, ces États s'engagent d'une manière déterminée et irréversible vers la sortie des énergies fossiles. Les énergies fossiles, pardonnez-moi de le rappeler,

Chacun n'emprunte peut-être pas les mêmes chemins, les mêmes outils, les mêmes modalités, mais nous sommes tous déterminés à laisser les énergies fossiles derrière nous. C'était, je crois, l'une de vos principales objections à l'adoption de ce texte, qui pose une interdiction une interdiction immédiate de délivrer de nouveaux permis d'exploitation des hydrocarbures sur le territoire national et des limites au renouvellement des concessions déjà acquises.

la France a rejoint la coalition pour la sortie du charbon, qui rassemble aujourd'hui plus de cinquante acteurs : des États, des villes, des entreprises et des investisseurs qui se désengagent du charbon.

mais aussi Quito et Cape Town, se sont engagées dans une déclaration à développer des zones « zéro émission » et à ne plus acheter que des bus à zéro émission à partir de 2025. Qu'on le veuille ou non, la fin des énergies fossiles est en train de s'écrire sous nos yeux. Mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi

La première assume le choix fait par le Gouvernement d'engager une transformation irréversible de notre modèle énergétique pour retrouver une forme de souveraineté dans ce domaine. La seconde, que vous avez défendue,

portaient atteinte à la cohérence du texte, à son ambition et au souhait du Gouvernement d'introduire dans notre droit les principales conséquences de l'accord de Paris, Comme l'a déclaré le Président de la République lors du sommet du 12 décembre, gardons à l'esprit que, en l'état, nous sommes en train de perdre la bataille climatique. Dès lors, nous avons le choix entre céder à une forme de

je vous invite à poursuivre sereinement nos échanges, à débattre des ultimes améliorations que nous pourrions apporter à ce texte. Nous le faisons sous le regard de nos concitoyens. Je sais que le Parlement a toujours fait a toujours fait preuve de responsabilité sur les questions environnementales. Un certain nombre de lois ont été votées dans une forme de magnifique consensus. C'est ainsi sous votre impulsion qu'a été

à poursuivre nos échanges, pour faire entrer l'accord de Paris dans notre droit et pour écrire ensemble une nouvelle page de la lutte contre le changement climatique. La parole

Madame la présidente, monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, alors que la position du Sénat a souvent été caricaturée, ce que je regrette vivement, car c'est très injuste, je tiens à redire l'état d'esprit dans lequel nous avions choisi d'aborder ce texte en première lecture. Dès lors que nous ne partageons pas l'approche du Gouvernement consistant à interdire une production nationale très résiduelle plutôt que plutôt que d'agir résolument sur la consommation, nous aurions pu, en effet, nous opposer frontalement et rejeter d'emblée le projet de loi qui nous était soumis. Au lieu de cela, et parce que l'enjeu climatique exige, au-delà des slogans et des symboles, une action collective efficace et déterminée, notre commission a dès l'origine cherché à améliorer le texte pour lutter véritablement contre le réchauffement planétaire. Le Gouvernement nous disait vouloir interdire la production d'hydrocarbures non pas pour elle-même, mais en raison de son effet sur le climat : nous l'avons donc pris au mot en confrontant les solutions proposées aux réalités du terrain. Car pour être irréversible, comme vous le souhaitez, monsieur le ministre d'État, l'évolution de notre modèle productif suppose d'être acceptable à la fois sur le plan économique et social. Au Sénat, nous n'oublions pas qu'un développement durable doit impérativement reposer sur trois piliers : l'environnement, le social et l'économie ; et c'est bien cet équilibre que nous avions visé en première lecture. Nos détracteurs nous ont opposé qu'à prévoir trop de dérogations, quand bien même celles-ci seraient strictement encadrées et justifiées, nous aurions dénaturé le texte et affaibli la portée du signal politique. Il me semble au contraire qu'en préférant le symbole à l'efficacité, en rejetant par principe toutes nos propositions, le Gouvernement et sa majorité se sont enfermés dans une approche dogmatique qui manquera sa cible, en n'ayant aucun effet sur nos émissions de gaz à effet de serre. D'ailleurs, nous contestons à ce gouvernement et à cette majorité le monopole de la lutte contre le changement climatique. Oui, le Sénat est plus que jamais déterminé à agir pour le climat. Oui, nous continuerons, pour cette raison, à défendre très concrètement la place du nucléaire dans le mix électrique, à plaider pour une tarification forte du carbone, à soutenir le déploiement des énergies renouvelables au meilleur coût pour la collectivité, ou à faciliter le développement maîtrisé de l'autoconsommation. Non, il n'y aurait pas d'un côté les vertueux, adeptes d'un « nouveau monde », et de l'autre les rétrogrades enfermés, pour citer le rapporteur de l'Assemblée nationale, dans « une vision défensive et passéiste de la transition écologique pour notre pays et notre tissu industriel Non, le Sénat n'a pas amendé le projet de loi parce que les sénateurs auraient « manifesté une incompréhension préoccupante des objectifs comme de la portée [du] texte ». En d'autres termes, dans l'esprit du Gouvernement et de sa majorité, il était impossible pour le Sénat d'adhérer à l'objectif tout en proposant une autre marche à suivre, sauf à ce que nous ayons tout simplement mal compris En l'état, ce projet de loi n'aura d'autre effet que de mettre fin au « produire en France », en dégradant à la fois notre balance commerciale et notre bilan carbone, et dans l'espoir d'un improbable signal envoyé au monde. À l'opposé d'une telle approche, le Sénat a défendu une autre vision, pragmatique et ambitieuse, qui développe nos filières industrielles, tout en accompagnant leur mutation pour réduire nos émissions. C'était le sens, en particulier, des dérogations que nous avions créées ou étendues en faveur des hydrocarbures à usage non énergétique, des productions connexes ou de la recherche. C'est ce même pragmatisme qui nous avait conduits à autoriser les régions d'outre-mer à exercer la compétence qui leur est théoriquement dévolue pour exploiter les ressources présentes au large de leurs côtes, et contribuer ainsi à leur développement économique et social. C'est enfin pour faire respecter la parole de l'État que nous avions souhaité un traitement moins brutal des demandes en cours d'instruction, et pour assurer un profit minimal aux exploitants que nous avions amendé l'encadrement du droit de suite. Aucun de ces apports majeurs n'a survécu en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale qui, à quelques modifications rédactionnelles ou exceptions près sur des sujets secondaires, a rétabli le texte issu de ses travaux en première lecture sur le volet « hydrocarbures Seul changement notable par rapport à cette version, l'adoption d'une définition nouvelle des techniques dites « non conventionnelles » posera sans doute des difficultés d'interprétation qui pourraient remettre en cause des méthodes autorisées jusqu'à présent. Au-delà des hydrocarbures, le projet de loi comportait une série de dispositions plus techniques sur lesquelles une grande partie, voire la quasi-totalité, des apports du Sénat a en revanche été conservée, notamment pour réformer le stockage souterrain de gaz naturel, conforter le régime d'indemnisation des producteurs d'énergies marines renouvelables en cas d'indisponibilité du raccordement, mieux encadrer la notion nouvelle de réseaux intérieurs, protéger les filières française et européenne de biocarburants contre la concurrence déloyale de produits importés, permettre aux communes de déployer des stations de recharge en gaz ou en hydrogène, réformer les sanctions applicables en cas de non-respect de l'obligation de pavillon français ou assouplir les obligations d'économies d'énergie des distributeurs de fioul domestique. Sur cet autre volet, je regretterai simplement le rétablissement de l'obligation de double distribution dans chaque station-service qui mettrait à la vente de nouveaux biocarburants, obligation que n'exige pas le droit européen et qui fragilisera encore un secteur de la distribution de carburants déjà sinistré. J'ajoute que l'introduction, à ce stade de la navette, d'une disposition nouvelle pour réduire les coûts de raccordement des méthaniseurs aux réseaux de transport est certes bienvenue sur le fond, mais méconnaît certainement la « règle de l'entonnoir » Au sortir de la nouvelle lecture du projet de loi à l'Assemblée nationale, le bilan apparaît donc très contrasté : sur le volet le plus politique du texte, c'est-à-dire sur les hydrocarbures, les députés n'auront fait droit à aucun de nos arguments. À l'opposé, sur les parties plus techniques, l'essentiel de nos apports aura été préservé, signe que la qualité de nos travaux, au moins sur ce plan, aura été reconnue. Mais dès lors que le Gouvernement et sa majorité jugent les fondements de leur texte « incontestables », il n'y a plus de place pour le dialogue entre nos deux assemblées, et rien n'indique qu'un nouvel examen des articles nous permettrait de progresser sur la voie d'un improbable compromis, ce qui justifie pleinement l'adoption d'une motion tendant À ceux qui, parmi vous, regrettent qu'une telle procédure écourte nos débats, je rappellerai que, malgré des délais très contraints, la première lecture avait été l'occasion d'un travail de fond qui avait permis, aux uns et aux autres, de faire valoir leurs positions, ainsi qu'en témoignent les très nombreux amendements présentés ou adoptés. S'il en était encore besoin, nos échanges de la semaine dernière en commission ont confirmé que les points de désaccord se sont cristallisés et qu'il sera difficile, sinon impossible, de faire encore évoluer le texte. Lors de cette réunion de commission, certains d'entre vous ont aussi fait part de leurs regrets de ne pouvoir parvenir à un consensus sur des sujets aussi primordiaux. Je fais mienne cette déception et je le dis d'autant plus que, sans trahir de secret, nous étions prêts à faire un certain nombre de concessions, y compris sur des sujets qui nous tenaient particulièrement à coeur, pour parvenir à un accord en commission mixte paritaire. malgré la qualité du dialogue noué avec les rapporteurs de l'Assemblée nationale, ces tentatives de conciliation n'auront trouvé, auprès de ces derniers ou du cabinet du ministre, aucun écho favorable. Il n'y avait donc aucun espace de négociation, sauf à renier la totalité de nos positions, et nous n'avons par conséquent plus d'autre choix que de rejeter l'ensemble du projet de loi. La parole

dans lequel nous nous sommes investis positivement, tant le symbole nous semblait important. Malheureusement, si le texte venant de l'Assemblée nationale comportait certaines failles, nos travaux les ont accentuées, réduisant quasi à néant les ambitions de ce projet de loi en laissant bien trop de place aux intérêts partisans et financiers des industriels pétroliers et gaziers, qui vont à l'encontre de l'intérêt général et environnemental. Bien naturellement, les députés ont rétabli leur texte, avec quelques évolutions notables et favorables, notamment la définition de la fracturation qui permet concrètement, à notre sens, que soit interdite l'exploitation des gaz et hydrocarbures de roche. Aujourd'hui, la nouvelle lecture va être courte, puisqu'une motion est déposée. Nous ne partageons ni cette démarche qui prive le Sénat de ses prérogatives ni les attendus qui nous semblent en décalage absolu avec l'urgence environnementale. Que dire de ce projet de loi en fin de parcours ? Si nous adhérons au symbole, nous aurions aimé qu'il aille plus loin, et ce de plusieurs manières. Tout d'abord, en plaçant à plus brève échéance la fin des permis de recherche et concession. 2040 nous semble bien lointain au regard de l'urgence climatique. Ensuite, parce que le droit de suite est maintenu, alors qu'il porte atteinte à la capacité de la puissance publique de maîtriser son mix énergétique et de définir sa politique minière. En outre, l'introduction de la notion de l'équilibre économique est une épine dans le principe même de l'arrêt de l'exploitation et de la recherche. Enfin, parce que ce texte n'envisage l'économie des énergies fossiles que sous le prisme de l'exploitation. Il fait l'impasse sur la définition d'une stratégie nationale en matière d'importation, et ne fixe aucune règle nouvelle sur le financement, y compris public, des activités d'exploitation des hydrocarbures à l'étranger. Or nous savons que ces questions sont importantes.

avec les avantages juridiques et fiscaux qui vont avec. En vertu de cet accord, la France ne pourra plus s'opposer à l'importation de sables bitumineux du Canada. Pour ne prendre que quelques exemples, cet accord entraînera une hausse des échanges entraînant à son tour une hausse des émissions de gaz à effet de serre, et mettra à mal le principe de précaution.

sur la COP23 la semaine dernière. Nous continuons donc, je le répète, de défendre l'idée d'un référendum, pour donner la parole au peuple qui va à l'encontre de l'objectif de ce projet de loi. Par ailleurs, le rapport d'Attac a également mis en lumière l'aide apportée par les banques nationales et les institutions financières publiques aux projets concernant les énergies fossiles. Ainsi, les banques françaises ont investi 844 millions d'euros dans les énergies fossiles depuis 2015, alors même que les énergies renouvelables ont vu leur financement baisser de 23 % au niveau mondial. La loi de finances pour 2018 continue une politique fiscale avantageuse de niches pour les énergies fossiles, qui coûteront la bagatelle de 7 milliards d'euros au budget national ! Nous ne pouvons plus continuer ainsi à manier le double discours, comme encore récemment lors du Derrière les promesses de décarbonation de l'économie, la réalité est tout autre. Après trois années de stagnation, les émissions humaines de dioxyde de carbone sont reparties à la hausse en 2017. C'est le constat des travaux publiés, le 13 novembre dernier, par par 15 000 scientifiques de 184 pays. Cette tribune enjoint aux responsables politiques que nous sommes de tout mettre en oeuvre pour « freiner la destruction de l'environnement » et éviter que ne s'aggrave l'épuisement des ressources que l'humanité tire de la planète. Le point de non-retour est presque atteint. Monsieur le ministre d'État, au-delà des symboles, la transition énergétique et écologique doit donc s'incarner. Plus un euro ne doit financer les énergies fossiles Par ailleurs, pour engager ce changement de paradigme, les transformations doivent être accompagnées et préparées. Le changement climatique, s'il est réfléchi et préparé, ne menace pas les emplois, comme je l'ai entendu, au contraire d'en créer. Ainsi, la plateforme emplois-climat indique qu'un million d'emplois seraient créés si nous investissions dans la transition énergétique. Il faut veiller à ce que les salariés des filières menacées aient le temps et les moyens de se reconvertir, mais il faut aussi préparer l'avenir, c'est-à-dire la protection de notre planète, de la biodiversité, qui est la condition même de la vie. Nous prônons, vous le savez, un pôle public de l'énergie, dégagé des impératifs de rentabilité et du marché, afin que notre pays se donne démocratiquement les outils pour favoriser les coopérations et la montée en puissance des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Ce pôle aurait pour mission de garantir pour toutes et tous un droit à l'énergie dans des conditions économiquement acceptables. Il est clair qu'aujourd'hui aucune énergie renouvelable n'est en capacité de répondre aux besoins de la consommation nationale. Pour autant, la question du produire mieux et plus et, en même temps, du consommer moins est donc centrale, tout comme celle de l'indépendance énergétique. Pour conclure, toutes ces questions doivent être débattues au sein de ce pôle public, qui devra avoir les moyens de mener cette politique audacieuse. Pour cela deux solutions

Madame la présidente, monsieur le ministre d'État, madame la rapporteur, mes chers collègues, nous abordons à nouveau ce projet de loi qui est l'une des premières mises en oeuvre de l'accord de Paris sur le climat, affichant les ambitions de la France et des cosignataires de réussir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, ambitions que je partage. Puisque la COP21 qui a entériné ce traité international a eu lieu en France, puisque la France s'est toujours montrée à l'avant-garde des défis planétaires et universels, il est légitime que la France soit l'un des premiers pays à se montrer exemplaire. Je souhaite vous le réaffirmer clairement, monsieur le ministre d'État : le groupe Union Centriste partage les objectifs environnementaux et de lutte contre le réchauffement climatique. Nous serons présents pour soutenir la politique énergétique de la France visant à réduire la consommation des énergies fossiles, qui permettra, entre autres, de contenir l'augmentation de la température en deçà de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et à tendre vers un objectif de 1,5°C. Nous saluons les Nous saluons les efforts que le Gouvernement entend mener dans les énergies renouvelables, qui seront utiles pour décarboner l'économie et la production énergétique. L'annonce de l'augmentation de 1 gigawatt des appels d'offres solaires par l'État et, surtout, le plan dévoilé par EDF visant à développer 30 gigawatts de solaire photovoltaïque entre 2020 et 2035 inscrivent la France dans ses ambitions de transition énergétique. Toutefois, monsieur le ministre d'État, il faudra être beaucoup plus offensif dans la réduction de la consommation. J'espère que l'État affiche la même volonté dans l'éolien, la géothermie, la méthanisation et dans le contenu de ses futurs contrats de transition écologique et solidaire à destination des territoires. Je connais des communes de mon département qui sont intéressées pour déployer ces énergies.

Je commence à avoir une certaine expérience et j'ai participé à quelques commissions mixtes paritaires dans ma vie parlementaire. Certaines étaient rudes, les convictions s'affrontaient et les débats rapprochaient les points de vue. Ainsi, bien souvent, les députés et les sénateurs arrivaient à un accord, parfois largement, parfois, mais les uns reconnaissaient les arguments et les expériences des autres. Or ce n'est pas ce que nous avons vécu le 21 novembre dernier ! Absolument ! Les nouveaux députés qui, paraît-il, s'inspirent de nouvelles méthodes de management et de démocratie participative, avec une volonté de bienveillance, ont dû oublier leur guide et leur manuel au Palais-Bourbon J'en profite pour saluer le travail de notre rapporteur, Élisabeth Lamure, qui avait apporté pour la majorité sénatoriale des ajustements sans détricoter le texte. Je suis certaine que d'autres mesures auraient pu être conservées par l'Assemblée nationale, dans un souci d'équilibre afin de lutter contre le dérèglement climatique.

malgré nos investissements en matière de transition énergétique, malgré le développement des énergies renouvelables- solaire, éolien, méthanisation ... -, nous ne serons pas totalement sortis de l'ère des hydrocarbures. Nous en utiliserons beaucoup moins, mais nous en utiliserons encore ! Il est des secteurs où les palliatifs n'ont pas encore été trouvés. En aviation, par exemple, il n'y a pas d'alternative au kérosène. En 2040, il est donc vraisemblable que nous continuions à utiliser des hydrocarbures, les techniques évoluant, mais pas aussi vite que nous l'imaginons. La question qui me fait douter de la pleine efficacité de ce projet de loi est celle-ci pourquoi importer des hydrocarbures, car nous y serons contraints, qui ont un impact carbone beaucoup plus fort que les hydrocarbures nationaux ? Ce projet de loi a pour objectif principal d'arrêter la recherche et l'exploitation des hydrocarbures en France, pas d'arrêter leur consommation. Vous ne proposez pas la fin des énergies fossiles, mais la fin du « produire en France » ! Sur un plan environnemental, le pétrole produit en France permet d'éviter l'émission de 100 000 tonnes de CO2 du fait de l'absence de transport. De plus, en se privant de la production nationale, la France favorisera plus encore l'importation de pétrole étranger pour lequel nous ne connaissons pas les conditions environnementales et sociétales d'extraction. En France, nous bénéficions d'un arsenal de normes et de contraintes permettant de protéger la biodiversité ou les sols. Il sera d'ailleurs intéressant de faire le bilan pour le climat, monsieur le ministre Nous consommerons toujours des hydrocarbures ; nous en consommerons véritablement moins, mais absolument importés ! Bref, vous maintenez malgré tout le cap de 2040. Les impacts se feront peut-être sentir au plan écologique, mais ils se feront assurément sentir au détriment des territoires Ces concessions structurent des bassins de vie de nos départements. Il ne faut pas oublier que ces exploitations engendrent des revenus financiers importants pour les collectivités. Dans la Marne, nous avons des idées, mais aussi un peu de pétrole, et les ressources de la redevance communale et départementale des mines représentent 1,8 million d'euros. On pourrait additionner ainsi l'ensemble des départements impactés par cette législation outre, ces installations sont de véritables écosystèmes industriels qui bien souvent se situent dans des zones déjà touchées par la crise économique ou éloignées des zones d'emplois dynamiques, qui drainent des centaines d'emplois directs et indirects. C'est pourquoi, monsieur le ministre d'État, il faut étudier la possibilité de créer un fonds permettant d'accompagner économiquement les territoires pénalisés par la fermeture de sites liée à la fin de l'exploitation des hydrocarbures. Ces fermetures peuvent avoir des conséquences économiques et sociales graves. Ne pouvant créer ce fonds par voie d'amendement, je propose la remise d'un rapport dans un délai assez bref, afin de rassurer l'ensemble des acteurs- élus, entreprises et salariés -touchés sur le terrain. Convaincue que notre pays devra toujours importer des hydrocarbures pour poursuivre ses activités, je propose que ce fonds soit utilement alimenté par une taxation des importations d'hydrocarbures. Ainsi, il pourrait être créé une forme de cercle vertueux entre ces importations et la revitalisation des territoires. C'est un point important pour le développement économique dans le monde rural qui a finalement été assez peu débattu. Je vous remercie, monsieur le ministre d'État, d'être attentif à l'avenir de nos territoires et à la solidarité pour la transformation de ceux-ci. Le dispositif que je propose répond à ces objectifs et à notre ambition partagée. J'insiste enfin : le groupe Union Centriste considère la transition énergétique et écologique comme un besoin vital, crucial. Je ne sais pas si ce texte sera utile, mais ce qui est certain, c'est que personne ne détient seul la vérité : les députés de la majorité présidentielle devraient le prendre en compte ! La parole

Voilà un texte qui aurait mérité autre chose que la procédure accélérée qui est imposée au Parlement. Voilà un texte qui aurait également mérité plus de volonté- de part et d'autre -dans l'objectif de parvenir à un consensus, par plus d'échange, plus de dialogue et plus de désir d'aboutir à un texte coconstruit entre députés et sénateurs.

Nous devrions unanimement cesser de douter, de tergiverser et de reporter certaines décisions. Nous devrions plutôt unir nos forces dans cette lutte contre le chamboulement climatique. Force est de constater que ce n'est pas encore le cas, vu l'état des discussions, sur ce texte notamment. Or faut-il insister, encore et encore, quitte à se répéter, sur la vulnérabilité des sociétés humaines devant les forces de la nature lorsque ces sociétés sont construites dans le déni de l'environnement ? Faut-il rappeler que nous risquons de perdre cette bataille contre le changement climatique ? Faut-il rappeler toujours et encore qu'il est urgent de passer d'une société fondée sur une consommation abondante d'énergies fossiles à une société plus sobre et écologiquement plus responsable ? C'est tout l'enjeu de la transition énergétique. C'est tout l'enjeu de la COP21 et de l'accord de Paris. C'est tout l'enjeu du présent texte, qui vise à envoyer un signal fort au monde entier, comme la France a su en envoyer dans son histoire, en faisant de notre pays le premier pays au monde à laisser les hydrocarbures dans le sous-sol.

Les ruptures dans nos comportements se confirment, certes trop lentement encore. L'État, les collectivités territoriales, l'économie sociale et solidaire se mettent en mouvement. Le verdissement de l'économie française est certain, même si les résultats sont encore contrastés. Avec ce projet de loi, tel que modifié en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, la France s'engage résolument dans un développement post-pétrolier, réellement durable, en commençant par se libérer des énergies fossiles une brique de plus en matière de lutte contre le chamboulement climatique ou, dit autrement, une impulsion supplémentaire sur un mouvement engagé depuis quelques années et qui se doit de devenir irréversible. Cela dit, je voudrais insister sur les quatre corollaires qui doivent impérativement découler de la mise en oeuvre de ce projet de loi. l'indispensable et urgente modification de nos comportements et de nos modes de consommation, ce qui implique une véritable transformation culturelle en ce domaine. Deuxièmement, la réduction de nos consommations d'énergies fossiles. le développement des énergies renouvelables, encore entravées par certains blocages administratifs et par des processus décisionnels complexes. Quatrièmement, enfin, un investissement massif dans la recherche et la formation l'objectif étant de construire un nouveau modèle économique nous permettant d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. La loi de transition énergétique de 2015 et le texte que vous nous présentez, monsieur le ministre d'État, constituent les premières briques de l'édifice à construire. Or certaines des modifications introduites par le Sénat en première lecture nous paraissent de nature à compromettre l'irréversibilité des mesures permettant de lutter contre le changement climatique en vidant de son sens l'essentiel du projet de loi. Ce fut un mauvais signal donné par la majorité sénatoriale, qui expliqua que le groupe socialiste et républicain ait pu voter contre ce texte. Certes, le Sénat avait apporté un certain nombre de compléments utiles sur des dispositions techniques, notamment aux articles 5 , 5 , 5 A, à l'article 4 relatif au stockage du gaz ou encore à l'article 11 sur les certificats d'économie d'énergie pour les petites entreprises de fioul, mesure chère à Martial Bourquin et à Angèle Préville, ici présents. tout aussi objectivement, on ne pouvait que déplorer le détricotage qui eut lieu avec la multiplication des dérogations, des exceptions ou des assouplissements terme « dérogation » était devenu le maître mot du texte élaboré par la majorité sénatoriale. Ces dérogations faisaient perdre tout son sens à ce texte en le dénaturant et en en brouillant le signal. Je ne les cite pas, chacun ici les connaît, mais elles furent autant de contresens regrettables, qui m'ont fait dire une fois de plus que le signal donné par le Sénat n'était pas bon du tout. et républicain a donc fait connaître son désaccord avec la majorité sénatoriale. Pourtant, très sincèrement, j'avais un temps espéré qu'il pourrait y avoir un consensus national concernant la transition énergétique et la sortie des énergies fossiles, ... Nous aussi ! ... donc que nous pourrions aboutir à un compromis en matière de lutte contre le changement climatique. Je pensais naïvement qu'après la Charte de l'environnement inscrivant le principe de précaution dans la Constitution sous Chirac, après le Grenelle de l'environnement sous Sarkozy, après la loi de transition énergétique de 2015, le succès de la COP21 et de l'accord de Paris sous Hollande, nous pouvions sous Macron, ici, au Sénat, une majorité d'idées en faveur de la sortie des énergies fossiles. C'était erreur ! Certes, sur les principes, tout le monde est d'accord, mais sur les principes seulement. Or, face au dérèglement climatique,

car notre ligne doit être claire et dépourvue d'ambiguïté. Ce texte est loin de se réduire à un symbole. D'ailleurs, s'il n'avait été que symbolique, comme certains l'affirment, et s'il n'avait été qu'une coquille vide, comme d'autres l'ont laissé entendre, pourquoi la majorité sénatoriale l'aurait-elle vidé de sa portée et de son sens en de nombreux points ? Gardons-nous d'oublier, mes chers collègues, que l'objectif de l'accord de Paris est bien de sortir des énergies fossiles. Ce texte prévoit d'organiser cette sortie de manière progressive, en douceur, sur deux décennies, mais fermement et de manière irréversible. Ce texte doit être effectivement le symbole d'une France qui tient ses engagements dans son combat contre le dérèglement climatique, qui reste à l'avant-garde en ce domaine, et donc en situation d'entraîner d'autres pays dans la seule voie qui vaille, celle de la neutralité carbone. Bref, nous approuvons le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale et nous soutenons votre action en ce domaine, monsieur le ministre Il est vraiment dommage que la commission des affaires économiques ait proposé d'évacuer ce texte au travers de la question préalable, nous empêchant ainsi de le retravailler et de nous donner une chance, aussi petite soit-elle, d'aboutir, par une majorité d'idées, à un texte consensuel.

Madame la présidente, monsieur le ministre d'État, madame la rapporteur, mes chers collègues, l'échec de la commission mixte paritaire nous conduit à nous exprimer une seconde fois sur ce projet de loi mettant fin à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures.

L'urgence à agir fait l'unanimité parmi la communauté scientifique. Je pense encore à l'appel des 15 000 experts mondiaux à la une du journal voilà quelques jours. Cela a été dit à plusieurs reprises en première lecture : notre planète se meurt ... La dernière fois que la Terre a connu de telles teneurs en CO2, c'était il y a 3 ou 5 millions d'années. Des efforts ont été entrepris depuis plusieurs années, mais les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont évidemment insuffisants pour tenir le cap de la limitation de l'augmentation des températures d'ici à 2100. Face à ce constat terrible, les velléités de certains dirigeants étrangers freinent l'engagement international à lutter contre le changement climatique. L'ombre de l'échec du protocole de Kyoto plane sur l'accord de Paris. L'agrégat des engagements internationaux nous inscrit aujourd'hui dans une trajectoire d'élévation de En outre, l'annonce du président Trump résonne encore comme un coup de semonce terrible dans le ciel des relations internationales. Pour autant, nous ne pouvons pas nous résoudre à baisser les bras. Tout au contraire, cet isolationnisme américain, qui n'est pas aussi total qu'on le croit- Dieu soit loué ! -, doit nous conduire à porter internationalement le flambeau du développement durable. Le président Chirac avait été l'un des premiers à le dire au début des années deux mille, à Johannesburg, faisant de la France un acteur primordial de la protection de l'environnement. de cet héritage et de mener l'engagement international à préserver la planète. Le Président de la République veut, avec vous, monsieur le ministre d'État, faire de la France un chef de file de la lutte contre le changement climatique. Nous éprouvons une grande fierté à soutenir cet engagement. était l'objectif de sa déclaration de l'été dernier : ! Oui, faisons de cette planète un endroit meilleur. Ce projet de loi est la première pierre de cet édifice. Le Président l'a posée. À nous, parlementaires, d'y apposer le ciment nécessaire pour renforcer cette structure et en faire une fondation durable de notre politique environnementale.

d'échanger avec vos collègues ministres à Bercy pour que le projet de budget pour 2019 intègre le respect des objectifs du développement durable dans les bleus budgétaires de l'administration.

pour parvenir à un texte adoptable et responsable. Cela n'a pas été le cas, et nous le regrettons. De manière générale, notre groupe veut cesser d'opposer écologie et économie. Le ministre de la transition

pour notre planète est bon pour notre économie ! Si les engagements que nous prenons aujourd'hui nous paraissent coûteux, voire douloureux pour certains, ils

ce puissant et symbolique message de la France pour concrétiser l'accord de Paris. Il ne s'agissait pas de résoudre tous les problèmes, mais d'envoyer un message au monde.

Nous avons largement débattu de ce projet de loi en première lecture, notamment de sa portée « symbolique », puisque 1 % seulement des hydrocarbures consommés en France sont extraits sur le territoire. Cette loi son véritable sens si on la considère comme le point de départ d'une véritable transition énergétique. Il faut abandonner les énergies fossiles, décarboner notre économie, investir massivement dans les énergies renouvelables et dans les économies d'énergie, opérer la

Nous devons aussi progresser sur les agrocarburants, afin que le changement d'affectation des sols, y compris indirect, soit pris en compte dans l'évaluation du bilan environnemental. Nous devons absolument laisser 80 % des réserves d'hydrocarbures dans le sous-sol si nous voulons avoir une chance d'éviter la catastrophe climatique. La France doit montrer l'exemple et doit en être fière. Nous pouvons être leaders dans la lutte contre le bouleversement climatique. Ne laissons pas passer cette opportunité Si le Sénat, en première lecture, a contribué à enrichir ce texte en consolidant des mécanismes essentiels pour la transition,

permettent à tous les exploitants de poursuivre l'extraction, notamment à travers le renforcement du droit de suite, inscrit dans le code minier, mais aussi avec la possibilité offerte aux exploitants de gisements de demander des dérogations allant 2040 afin d'assurer « une rémunération normale des capitaux immobilisés compte tenu des risques inhérents à ces activités ». C'est l'un des éléments de dérégulation incompréhensibles issus des discussions au Sénat. L'Assemblée nationale est évidemment revenue à un texte

de l'examen du texte dans le détail, ce que nous regrettons vivement ! Ce projet de loi est le premier marqueur de la politique de transition que vous avez voulue, monsieur le ministre Bien au-delà du symbole, c'est un signal fort adressé à la suite de sommets mondiaux de plus en plus alarmistes quant à notre capacité à réagir. C'est aussi un texte qui donne sa vraie place au politique face aux intérêts économiques et financiers. La majorité sénatoriale a remanié le texte à la grande satisfaction des industriels du secteur pétrolier et gazier. La question de l'urgence climatique se pose pourtant comme une priorité essentielle tout récemment, le climatologue Jean Jouzel a affirmé qu'il ne nous restait que trois ans pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre et espérer rester en dessous de la barre des 2°C. Nous aurons des positions

pour diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre en Europe, mais aussi dégonfler la bulle financière et créer plus de 5 millions d'emplois à l'échelle européenne,

bon nombre de parlementaires, toutes formations politiques confondues, ont participé il y a quelques jours au, dans une démarche d'adhésion totale. L'une des tables rondes organisées avait pour titre : « Renforcer les politiques publiques pour la transition écologique et solidaire. Chacun convient en effet que les gouvernements doivent jouer le rôle de garant des objectifs de l'accord de Paris. Si la mobilisation de tous est nécessaire pour atteindre nos objectifs, les politiques publiques doivent accompagner et envoyer des signaux forts pour que l'ensemble des acteurs puissent transformer leurs modes de production et de consommation vers des solutions bas carbone. À la lumière des impacts déjà ressentis du dérèglement climatique, il est indispensable de renforcer la résilience et l'adaptation pour protéger encore davantage les citoyens des événements climatiques extrêmes. Les politiques publiques doivent intégrer l'horizon de long terme en fixant, par exemple, des objectifs de neutralité carbone. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, leur donner un prix est indispensable. Enfin, la résilience et la capacité de nos infrastructures à faire face aux chocs liés au dérèglement climatique doivent être au coeur des préoccupations. À ce titre, le gouvernement français s'est pleinement saisi du sujet et accélère la transition énergétique pour faire de l'accord de Paris une réalité pour tous les Français. Oui, le changement climatique nous impose de nous rassembler, au-delà de toutes les barrières politiques, culturelles et sociales, pour faire face à cet enjeu. Nous nous devons de sceller cette cause commune, car le changement climatique ne connaît ni frontières ni clivages politiques, et nous n'avons plus que quelques années pour inverser la tendance. Nous avons encore les moyens d'éviter le pire, mais cela demande une action résolue, car nous entrons dans une phase décisive. La réponse doit être à la hauteur des enjeux. C'est dans cette optique qu'en novembre dernier, nous avons examiné un projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement. Je ne reviens pas sur les diverses mesures contenues dans ce projet de loi, qui ont donné lieu, dans notre assemblée, à moult débats en commission et en séance publique, permettant de mesurer les fractures qui n'ont rien d'hydraulique entre les uns et les autres, sur un sujet qui aurait sans doute mérité mieux que certains des arguments que nous avons pu entendre et qui donnaient parfois l'impression que nous étions revenus à l'époque de la révolution industrielle. Premier pays à traduire cet engagement dans une loi, la France peut se donner ainsi les moyens de sortir de manière irréversible de la production d'énergies fossiles. Fidèle à sa vocation universaliste, elle souhaite inciter les autres pays signataires de l'accord de Paris sur le climat à intensifier l'effort de lutte contre le réchauffement climatique. Si notre assemblée a apporté des améliorations d'ordre technique qui ont été préservées, il est profondément regrettable que la majorité sénatoriale ait dénaturé ce projet de loi en adoptant une position pour le moins anachronique. Alors que nous venons de vivre, la semaine dernière, quatre jours dédiés au climat avec comme point d'orgue le, qui vise à verdir la finance et à accélérer la mobilisation des moyens financiers publics et privés, alors que les progressistes du monde entier se sont réunis à Paris, je déplore que la majorité de notre assemblée ait soutenu une vision passéiste et rétrograde de ce que doit être la transition énergétique. Pourtant, le projet que vous avez présenté, monsieur le ministre d'État, est responsable, équilibré et porte l'ambition d'un texte fort, symbolique, engageant pour la France en matière de lutte contre le dérèglement climatique, tout en veillant à préserver nos territoires, nos entreprises et les sites industriels concernés et à les inscrire dans une vision d'avenir de la transition écologique et solidaire. Réunie le 21 novembre dernier, la commission mixte paritaire a échoué à trouver un terrain d'entente et je rejoins mes collègues députés qui ont indiqué que « les sénateurs ont manifesté une incompréhension préoccupante des objectifs comme de la portée du texte Sur un sujet qui concerne l'avenir de nos enfants et qui devrait être dénué de position idéologique, alors même qu'en 2002, au sommet de la Terre de Johannesburg, le président Jacques Chirac lançait une alerte climatique au monde en déclarant : « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs », la majorité sénatoriale a choisi de fermer les yeux. C'est une attitude dommageable, pour ne pas dire plus. Arguer que le Sénat a défendu « une vision différente, à la fois pragmatique et ambitieuse, qui entend permettre le développement, chaque fois que c'est possible, de nos filières industrielles tout en accompagnant leur mutation pour réduire nos émissions » est un non-sens. Vous entendre, madame la rapporteur, nous dire que « ce projet n'aura d'autre effet que de mettre fin au " produire en France " au prix d'une dégradation de notre balance commerciale et dans l'espoir d'un improbable signal envoyé au monde » est une aberration à nulle autre pareille. C'est la vérité, malheureusement ! Au lendemain de ce formidable sommet pour la planète, c'est une aberration politique qui montre à quel point notre assemblée peut être rétrograde et à rebours des défis de notre temps. Cette aberration donne un signe on ne peut plus mauvais à l'opinion française, mais aussi au-delà, sur la façon dont le Sénat entrevoit l'avenir de la planète et des générations futures. Oui, la portée de ce texte est d'abord et avant tout symbolique, mais chacun sait que l'on construit l'histoire avec des symboles. « Là où il y a une volonté, il y a un chemin », disait Lénine, pourtant peu connu pour son tropisme sur la préservation de notre écosystème. Il n'était pas le seul ! Quant au chemin, il reste celui des énergies fossiles et du, ce qui est un non-sens historique, une faute qui engage notre responsabilité collective et dont nous serons comptables, mes chers collègues. Monsieur le ministre d'État, vous avez récemment déclaré : « Les énergies fossiles appartiennent au modèle énergétique et économique du passé.

Madame la présidente, monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, le projet de loi mettant fin à la recherche et à l'exploitation d'hydrocarbures que nous examinons en nouvelle lecture aujourd'hui n'est pas très éloigné du texte qui nous a été soumis en première lecture. suite de l'échec de la commission mixte paritaire, l'Assemblée nationale a en effet rétabli, à quelques mots près, la rédaction issue de ses travaux sur le volet « hydrocarbures », qui constitue le coeur de ce projet de loi. Les députés n'ont pas tenu compte de nos critiques et des propositions que nous avions faites. Nous regrettons notamment qu'ils soient revenus sur une disposition introduite sur l'initiative de la commission des affaires économiques et de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, qui visait à sanctuariser les activités de recherche publique sur les hydrocarbures. À notre sens, l'arrêt progressif de la production d'hydrocarbures ne doit pas conduire à cesser toute recherche dans notre sous-sol. Continuer à investir dans la recherche et la connaissance de notre sous-sol est essentiel. Il nous paraissait nécessaire que cela soit inscrit clairement dans la loi. De même, la disposition que nous avions adoptée pour garantir aux entreprises la possibilité de poursuivre leurs activités après 2040 afin de rentabiliser leurs investissements de prospection et d'exploitation, tout en dégageant un profit raisonnable, n'a pas été retenue par l'Assemblée nationale. Nous relevons cependant que, sur les autres parties du texte, plus consensuelles, les députés ont conservé la plupart des apports techniques du Sénat. Nous pensons en particulier à l'extension de l'indemnisation des producteurs d'énergie éolienne maritime par le gestionnaire de réseau en cas d'avaries ou de dysfonctionnements, ou aux dispositions relatives à la qualité de l'air, sur lesquelles la commission de l'aménagement du territoire s'était saisie pour avis. Ces apports ne suffisent cependant pas à rendre possible l'adoption de ce projet de loi en l'état. Les lacunes du texte que nous avions dénoncées lors de l'examen en première lecture demeurent entières.

Mais tel n'est pas l'objet de ce texte, qui n'aura aucun effet sur notre consommation d'hydrocarbures, et donc sur nos émissions de CO2. Il ne répond aucunement aux objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre que notre pays s'est fixés dans le cadre de l'accord de Paris. Nous attendions plus du Gouvernement pour son premier texte en matière d'environnement et d'énergie ! Les mesures que contient ce projet de loi auraient dû être examinées dans le cadre d'un débat plus large sur la politique de transition énergétique à mener et sur l'évolution de notre mix énergétique à moyen et long terme. Elles auraient dû par conséquent s'accompagner de mesures relatives au développement des énergies renouvelables ou à la réduction de la consommation énergétique des particuliers et des entreprises pour former un « tout » cohérent. Nous regrettons qu'en matière de transition énergétique, des débats aient lieu de manière fragmentée, avec des annonces qui se succèdent sur la rénovation thermique des bâtiments, sur la hausse de la fiscalité carbone ou encore sur le report de l'objectif de baisse de la part du nucléaire dans la production électrique à 50 %, sans que l'on dispose d'une vision d'une vision globale sur la politique énergétique menée. Or la clé d'une transition énergétique réussie, c'est un cap politique clair, une réglementation simple et lisible et des financements ambitieux. Nous attendons donc du Gouvernement qu'il publie rapidement une nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie et qu'il prenne les mesures législatives, réglementaires et financières nécessaires pour favoriser la transition de notre modèle énergétique. Nous pensons en particulier aux mesures à prendre pour faciliter la création de parcs solaires et éoliens terrestres et maritimes, qui pâtissent aujourd'hui de délais beaucoup trop longs de mise en oeuvre. De même, nous regrettons que l'interdiction de la production d'hydrocarbures n'ait pas été assortie d'une réflexion sur la qualité de nos importations d'hydrocarbures et sur la possibilité de différencier les hydrocarbures importés en fonction de leur bilan carbone sur l'ensemble de leur cycle de vie. Avant de mettre fin à une production nationale d'hydrocarbures plus « propres » que les hydrocarbures importés, il aurait fallu se donner les moyens de substituer aux énergies fossiles des énergies moins carbonées. Préparé et adopté dans la précipitation, ce projet de loi n'a pas laissé suffisamment de temps aux acteurs concernés pour mener à bien toute cette réflexion. Bien sûr, le monde change Mais ne nous faites pas de procès d'intention et arrêtez de nous donner des leçons : nous partageons tous les mêmes objectifs, mais nous envisageons des voies différentes pour les atteindre. Monsieur le ministre d'État, il n'y a pas, d'un côté, les gentils, vertueux et éclairés que vous seriez et, de l'autre, les méchants, irresponsables et pollueurs que nous serions. Votre vision symbolique et notre vision réaliste auraient pu se retrouver, mais ce ne fut pas le cas en commission mixte paritaire face à l'intransigeance des députés incarnant le prétendu

chers collègues, essayons de tirer certains enseignements de la discussion qui nous réunit aujourd'hui à propos du projet de loi relatif à la fin de la recherche des hydrocarbures, sur fond de COP21 et, plus près de nous, de COP23. Chacun s'accorde à reconnaître que les énergies fossiles doivent être abandonnées et qu'elles doivent sortir autant que faire se peut de notre vie au quotidien. Ce texte a pour ambition de donner une crédibilité à notre pays sur la scène internationale en matière de lutte contre le changement climatique, l'effet de serre et les conséquences dramatiques des particules en termes de santé publique. L'objectif du Gouvernement, que nous partageons, est la neutralité carbone à l'horizon 2050. Si toutes les tendances politiques s'accordent sur cette ambition, les moyens sont contestés, comme viennent de le rappeler nos excellents collègues rapporteurs Élisabeth Lamure et Jean-Marc Boyer. Ainsi, les positions du Sénat et de l'Assemblée nationale sont très divergentes, en particulier sur la possibilité d'accorder des permis pour la recherche d'hydrocarbures. Je regrette vraiment l'échec malheureux de la commission mixte paritaire du 21 novembre, mais, dans le même temps, je me réjouis que l'Assemblée nationale et le Sénat aient conservé une disposition introduite par la Haute Assemblée, fruit d'un amendement que j'avais déposé avec plusieurs de mes collègues du groupe Les Républicains. Cette disposition a été adoptée conforme. Le projet de loi aura au moins permis d'évoquer l'avenir des biocarburants. Je salue la position du Gouvernement, qui a enfin suivi le Sénat dans sa sagesse en maintenant un amendement à l'article 6 concernant le contrôle de la qualité environnementale des biocarburants. Le Sénat a en effet alerté sur la concurrence déloyale que représentent, pour les filières de production européennes, les biocarburants importés de certains pays comme l'Argentine ou l'Indonésie, dont les exigences sont moindres. La disposition proposée ne modifie pas les règles applicables pour les biocarburants européens dans des installations mises en service sur le territoire de l'Union européenne : le relèvement du seuil de niveau minimum de réduction des gaz à effet de serre reste déterminé par une mise en service avant ou à compter du 5 octobre 2015. En revanche, elle recule cette date d'effet au 1 janvier 2008 pour les installations situées dans des pays tiers. Il est prévu que cette différence, applicable dès l'adoption de la loi, disparaisse le 30 juin 2019, le temps que le recours déposé par les producteurs européens une plainte antidumping auprès de l'Union européenne règle ce dossier. Cette disposition antidumping protège les filières françaises et européennes contre l'afflux massif de biocarburants, qui seraient moins contrôlés et seraient, en outre, subventionnés par ces mêmes pays.

L'amendement que j'ai présenté, avec plusieurs de mes collègues, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2017 propose d'octroyer l'exonération de la taxe sur les véhicules des sociétés, la TVS, pendant une période de douze trimestres aux véhicules roulant au superéthanol E85, dont les émissions après abattement de 40 % sont inférieures ou égales à 75 grammes de CO2 par kilomètre. Monsieur le ministre d'État, il est grand temps,

les véhicules hybrides dits de la même manière que pour le GPL ou le GNV. Le Gouvernement ne tient pas compte de ces arguments pourtant majeurs. La situation actuelle est parfaitement subjective et contraire aux engagements pris par la France en matière de réduction de CO2 et de particules. Monsieur le ministre d'État, on peut légitimement s'interroger. Pourquoi le Gouvernement souhaite-t-il développer l'usage des carburants vertueux, sans s'en donner les moyens ? Est-ce un voeu pieux ?

du budget pour 2018 aurait été faible par rapport au bénéfice et au retour attendus. Monsieur le ministre d'État, est-ce trop cher payé pour le cheminement vers l'utilisation des biocarburants

qu'en dépit de toutes les argumentations possibles sur les dangers de notre modèle actuel, la commission des affaires économiques ait pu persister dans la remise en cause des points essentiels du texte, alors que les sirènes de l'urgence climatique se font de plus en plus stridentes et que les phénomènes climatiques sèment, partout dans le monde, inquiétude et désolation. Pourtant, j'imagine que chacun, ici, sent bien que le temps joue contre nous, que l'urgence d'agir se fait de plus en plus pressante

c'est dommage ! J'ai reconnu, lors de la discussion générale, que le Sénat, en première lecture, avait apporté un certain nombre de compléments utiles sur des dispositions techniques importantes. j'ai également déploré un certain détricotage du texte de la part de la majorité sénatoriale avec la multiplication de dérogations et exceptions vidant de leur sens des dispositions majeures et dénaturant donc l'essentiel du projet de loi. Je l'ai déjà dit,

plutôt que de tenter d'évacuer ce texte par le biais d'une motion, aurait pu faire oeuvre utile, en essayant de rapprocher les points de vue, d'améliorer certaines dispositions et d'en corriger d'autres.

nous voulons que la France s'engage clairement dans la sortie des énergies fossiles et dans un développement économique post-pétrole, réellement durable, conformément à l'objectif de l'accord de Paris Pour cela, il faut que cette sortie soit irréversible et sans dérogation ou exception. Pour nous, il s'agit- et nous vous soutenons bien volontiers, monsieur le ministre d'État, dans votre action -d'atteindre le plus rapidement possible la neutralité carbone, en bornant ainsi le réchauffement climatique en dessous de 2°C. Nous persistons donc à dire que ce projet de loi doit être un texte de rupture, qui en finisse avec un certain laisser-faire consistant à reporter les décisions difficiles à plus tard, de préférence sur les générations futures Il n'est tout de même pas si difficile de reconnaître que notre modèle actuel n'est plus durable et que la trajectoire qui en résulte n'est plus soutenable, dès lors qu'elle conduit chaque jour connu ! Non seulement nous voulons que ce projet de loi conserve toute son ambition, mais nous persistons à dire qu'il doit aussi être responsable, non seulement en donnant- comme c'est le cas -de la visibilité aux entreprises et territoires impactés,

et entreprenant ! Bref, nous sommes convaincus que, face à l'urgence climatique, écologique et sociale, nous devons, ici et maintenant, nous engager en faveur d'une économie fondée sur un autre modèle, plus durable, plus juste et porteur de croissance et d'emplois. Cela passe

ne souhaiteraient pas, ensuite, exploiter. J'aurais aimé vous convaincre que la cohérence et l'exemplarité produisent des résultats et nous donnent une crédibilité et une capacité d'entraînement. Je n'ai pas réussi à vous convaincre et je regrette le choix de déposer cette motion- je le dis franchement -, d'autant que le Sénat

La transition écologique et solidaire que je défends, avec d'autres, a besoin de mutualiser toutes ces intelligences. C'est pourquoi je regrette franchement le dépôt de cette motion,

grande mutation, vous verrez qu'elle apportera beaucoup plus de bénéfices que de contrariétés ;, elle nous apportera de lourdes contrariétés, si à un moment ou à un autre, nous ne nous retrouvons pas sur l'essentiel. En tout cas, j'espère que, malgré votre opposition,

c'est l'une des qualités de ceux qui s'expriment dans cette enceinte ... Pourtant, devant l'enjeu, notre incompréhension sur l'essentiel et notre incapacité à la dépasser me plongent, comme M. le ministre d'État, dans une forme de tristesse. Je ne parviens pas à comprendre

plus opérationnel. Bien sûr, nous n'avons pas trouvé de position commune sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures, mais nous avons introduit de nouvelles dispositions, souvent pragmatiques

que très peu les effets de communication, mais que nous partageons avec vous, monsieur le ministre d'État, l'objectif ultime, celui de la protection de notre planète et de l'engagement pour le climat.

d'un glorieux sénateur qui a contribué à l'histoire de notre pays, Édouard Herriot : « La persévérance dans une idée juste en amène le succès tôt ou tard.

J'informe le Sénat que des candidatures ont été publiées pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte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 L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations

Madame la présidente, monsieur le rapporteur de la commission des lois, la proposition de loi en discussion aujourd'hui s'inscrit dans la continuité d'un travail législatif qui a considérablement occupé le Parlement ces dernières années- tous les sénateurs, que je salue, ici présents le savent -, celui de la répartition des compétences entre les différents niveaux de collectivités. Ce chantier a, pour ainsi dire, occupé le Parlement de manière quasi continue durant la précédente législature, accompagnant les mutations très profondes de l'organisation, des ressources et des missions des collectivités locales mutations institutionnelles, évidemment, chacun le sait, avec la création des grandes régions, la naissance de métropoles, l'émergence de communes nouvelles, l'affirmation de collectivités à statut particulier, telles que la métropole de Lyon, la Ville de Paris ou la collectivité de Corse, la rationalisation de la carte intercommunale ; mutations également des compétences exercées par les différents niveaux de collectivités. La simplification de la répartition des compétences a été de pair avec la révision de nos architectures institutionnelles.Pas un territoire n'a été exempt de ces évolutions. Tous ont été et sont encore concernés par cette question de la distribution des compétences entre les différents niveaux de collectivités.

Cette demande, le Gouvernement l'a entendue, comprise et faite sienne. Voilà les raisons pour lesquelles, comme le Président de la République l'a confirmé au congrès des maires le 23 novembre dernier, il n'y aura pas de nouvelle grande transformation institutionnelle pour les collectivités territoriales. Stabilité et continuité n'excluent cependant pas de procéder à des améliorations. Mettre en oeuvre la loi n'interdit pas non plus de l'accompagner, non seulement pour l'expliquer, mais aussi pour en corriger les imperfections, en résoudre les difficultés d'application. Le Gouvernement s'est donc engagé à accueillir favorablement de telles initiatives et à mettre à l'étude les améliorations qui paraîtraient possibles dans la répartition des compétences entre collectivités, après avoir pris le temps de la concertation. À la demande du Premier ministre, j'ai d'ailleurs été mandatée pour organiser ces concertations et en tirer, au nom du Gouvernement, les conclusions utiles. Avant d'évoquer la présente proposition de loi, qui concerne la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, je voudrais revenir sur le deuxième domaine où des travaux ont été engagés, celui de l'eau et de l'assainissement. Comme vous le savez, une initiative parlementaire va se concrétiser dès le début de l'année 2018. Comme vous le savez également, j'ai animé un groupe de travail composé de huit députés et de huit sénateurs. Ce groupe a procédé à de nombreuses auditions et examiné la nature des difficultés posées par la loi NOTRe, telle qu'elle existe actuellement. Je réunirai de nouveau ce groupe cette semaine pour examiner comment nos conclusions, qui sont unanimes, peuvent être transcrites dans un texte de loi.

Cette faculté sera ouverte pour le mandat en cours et pour le suivant. Deuxièmement, nous reviendrons sur les dispositions de la loi NOTRe qui avaient pour effet de procéder, trop fortement et de manière trop automatique, à la dissolution de syndicats de plein droit, en généralisant le principe de représentation-substitution des communes par les intercommunalités, y compris lorsque les syndicats regroupent deux EPCI seulement. Voilà ce que nous proposerons. Vous le voyez, nous n'avons pas hésité à rouvrir le débat de manière constructive pour trouver une solution qui satisfasse tout le monde, comme l'a indiqué le Premier ministre à Cahors. Je m'étais engagée à ce que ces travaux se fassent. Ils se font ! C'était un engagement du Gouvernement, confirmé par le Président de la République

simple : la gestion des cours d'eau et celle du risque d'inondation sont intimement liées. Telle est la raison pour laquelle le législateur a souhaité réunir dans une même compétence ces deux aspects. En outre, les risques d'inondation, comme les effets d'une dégradation des milieux aquatiques, ne connaissent pas de frontières. Ils menacent tous les territoires riverains des fleuves et cours d'eau, ceux situés en aval étant souvent plus exposés que ceux à l'amont. Voilà pourquoi le législateur a choisi d'organiser la solidarité territoriale en ces domaines, en confiant aux intercommunalités le soin d'exercer cette compétence. Il est évidemment question, en matière de GEMAPI, de solidarité entre les territoires. l'ai dit, la logique de la GEMAPI est donc une logique forte et de solidarité, mais sa mise en oeuvre s'est heurtée à quelques difficultés. Nos fleuves, rivières et ruisseaux ne sont pas toujours entretenus comme il le faudrait. De plus, la gestion des digues est assurément une compétence dispersée et pas toujours bien exercée. Ici, des digues appartiennent à des associations de propriétaires fragiles, qui n'assurent pas qui n'assurent pas bien leurs obligations d'entretien. Ailleurs, la propriété d'ouvrages anciens n'est pas bien définie. Là-bas, les collectivités n'ont pas su s'entendre et s'organiser pour mettre en place un système d'endiguement approprié. En d'autres endroits, l'État n'a pas toujours été un propriétaire prévoyant et diligent. Enfin, le législateur de 2014 n'a sans doute pas suffisamment pris le temps d'examiner ce qui pouvait déjà exister dans les territoires, avant même que la compétence GEMAPI ne voie le jour. effet, il est des territoires où des initiatives s'étaient structurées, parfois depuis longtemps, pour assurer l'entretien mutualisé des cours d'eau, au contraire d'autres territoires, où rien ne s'était fait. ne s'était fait. Dans des territoires très exposés à de violents risques d'inondations- je pense, par exemple, aux épisodes cévenols dans le Sud-Est -, des collectivités avaient pris des initiatives pour éviter que l'inertie ne cause, chaque année ou presque, des morts. Par ailleurs, à la suite de crises majeures de submersion marine, certaines collectivités s'étaient engagées dans des travaux ambitieux et au long cours, pour mieux protéger habitations et activités humaines. Or l'uniformité prévue par la loi MAPTAM avait pour effet d'empêcher ce type d'initiative, obligeant même à les déconstruire, dès lors qu'étaient concernées des collectivités autres que communales. C'était, chacun le sait et le mesure, une véritable difficulté pour ces territoires. Nous avons donc souhaité revisiter la compétence GEMAPI à l'aune de la philosophie de la Conférence nationale des territoires. Cette philosophie est simple, et le Premier ministre l'a parfaitement exprimée en ouvrant les discussions lors de la première réunion de la Conférence nationale des territoires au Sénat, le 17 juillet dernier : « En termes de compétences, nous voulons à la fois permettre aux libertés locales de s'exprimer, tout en conservant l'idée d'une stabilité globale du dispositif. Stabilité globale du dispositif », car il n'est pas question de remettre en chantier les équilibres qui viennent d'être trouvés. Je peux ainsi vous confirmer que le Gouvernement ne reviendra pas

Les intercommunalités exerceront donc la compétence GEMAPI à compter du 1 janvier 2018, une compétence qu'elles pourront, si elles le souhaitent, transférer à des syndicats d'un genre particulier : les EPTB et les EPAGE. Elles bénéficieront par ailleurs d'une nouvelle ressource fiscale pour leur permettre d'exercer cette compétence. Mais cette stabilité doit être assortie de conditions de mise en oeuvre de la loi qui permettent aux libertés locales de s'exprimer pleinement. Il apparaît en effet, dans le domaine de la GEMAPI, que la loi a conduit à certaines difficultés, parce que les règles qu'elle définit s'accommodent mal de la réalité et de la très grande diversité de nos territoires. Le Gouvernement a donc soutenu

affirmer clairement un principe de sécabilité des différentes composantes de la compétence GEMAPI, qui seul garantit aux collectivités territoriales leur libre organisation dans l'exercice de cette compétence. Mesdames, messieurs les sénateurs, cette

Des réponses devaient en effet être apportées à l'inquiétude des élus, qui se voient transférer des ouvrages et craignaient d'être immédiatement tenus responsables de leurs imperfections, de leurs fragilités, voire de leurs défaillances.

encore sur le signal très positif que constitue cette proposition de loi, à laquelle le Gouvernement est dans son ensemble très favorable. Ce texte matérialise en effet notre souhait d'adapter la loi, lorsque cela est nécessaire, pour permettre aux libertés locales de s'exprimer et pour tenir compte des initiatives prises par les collectivités territoriales et qui fonctionnent déjà, comme celles prises Il vient concrétiser les premiers engagements pris dans le cadre de la Conférence nationale des territoires et confirme que cet état d'esprit n'est pas que de façade : les engagements pris ont été tenus, et l'ont été rapidement. Je salue le travail législatif à la fois rapide et efficace qui a permis de susciter cette proposition de loi,

un référent, en l'occurrence l'intercommunalité, qui puisse faire oeuvre utile en assumant le chef de filat sur ces sujets. Forts de ces constatations, nous avons essayé

l'article 1 de la proposition de loi, qui permet aux départements et aux régions de poursuivre leur action en matière de GEMAPI au-delà

L'Assemblée nationale a entendu assouplir les modalités de transfert et de délégation de la compétence GEMAPI à un syndicat mixte, en prévoyant notamment la sécabilité interne des quatre missions constitutives de cette compétence, aux articles 1, 3 et 4. Si la commission des lois a émis de fortes réserves sur ce point,

a également maintenu la faculté dont disposent actuellement les EPCI à fiscalité propre de transférer leurs compétences à un syndicat sur une partie seulement de leur territoire, ou à plusieurs syndicats sur des parties distinctes de leur territoire, dans l'ensemble du champ de la politique

des gestionnaires d'ouvrages de protection contre les inondations prévu à l'article 1, au cas où un sinistre surviendrait pendant la période transitoire entre le moment de leur mise à disposition et celui de leur autorisation par le préfet. Elle a notamment étendu le bénéfice de ce régime de responsabilité limitée à l'ensemble des ouvrages de protection, et non aux seules digues, qui seraient mis à disposition du bloc communal par toute personne publique, et non par les seuls départements et régions. La commission des lois s'est également penchée sur la prévention des inondations et la maîtrise des eaux de ruissellement. Observant que de nombreuses et graves inondations étaient dues au ruissellement des eaux plutôt qu'à la crue d'un cours d'eau ou à une submersion, elle s'est interrogée sur l'opportunité d'élargir le périmètre de la compétence GEMAPI à la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, ainsi qu'à la lutte contre l'érosion des sols.

problématiques territoriales. Je forme donc à nouveau le voeu que, dans l'esprit des engagements pris jeudi dernier par le Premier ministre, nous puissions réellement prendre en compte les aspirations des acteurs des collectivités territoriales- et même, pourquoi pas, écouter la voix du Sénat ! La parole

des enjeux de sécurité et de santé considérables ont conduit le législateur à mettre fin à l'émiettement existant dans la gouvernance de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. C'est ainsi que, en 2014, la loi MAPTAM a confié aux EPCI à fiscalité propre l'exercice de la compétence GEMAPI à compter du 1 janvier 2016. loi avait pour ambition, simplement, de mieux structurer la maîtrise d'ouvrage à l'échelle nationale et de rationaliser l'organisation territoriale, marquée par l'enchevêtrement et la dispersion des pouvoirs locaux. Cette mesure fut à l'époque sans aucun doute trop hâtivement votée, sans aucune étude d'impact préalable sur les conséquences considérables qu'elle engendrerait. Aussi, sous la pression des élus locaux, la loi NOTRe a-t-elle repoussé de deux ans, au 1 janvier 2018, l'entrée en vigueur de la GEMAPI, faisant ainsi la preuve de l'imperfection de la loi de 2014.

Face aux inquiétudes légitimes et aux obstacles réels rencontrés sur le terrain, la proposition de loi que nous examinons cet après-midi vient très utilement répondre aux interrogations pratiques des élus locaux en clarifiant certains points et, en même temps, en assouplissant le dispositif. elle réaffirme le rôle des départements et des régions et précise le cadre de responsabilité des élus, même si nombre d'interrogations subsistent sur la capacité des maires à répondre de leur pouvoir de police. Elle assouplit aussi les modalités de transfert et de délégation de la compétence en élargissant la concertation entre les acteurs. Toutefois, certains élus regrettent qu'elle ne permette pas une discussion globale, appréhendant des missions connexes telles que les compétences « eau et assainissement », traitées dans le cadre d'une proposition de loi sénatoriale qui, bien que votée à la quasi-unanimité de notre assemblée, n'a pas été reprise à l'Assemblée Je salue, madame la ministre, votre volonté et celle du Gouvernement de trouver une issue positive à cette impasse. Vous le savez, nous serons très attentifs à vos propositions.

J'en salue l'esprit, qui fait confiance à l'intelligence territoriale pour définir l'échelon compétent par rapport aux particularités de chacun de nos territoires. Il est évident que, dans un territoire de montagne et un territoire côtier, les missions GEMAPI ne recouvrent ni les mêmes réalités ni la même ampleur.

cette réforme, louable, comporte un manque : son financement. Concrètement, elle plonge les élus locaux dans un dilemme : créer un nouvel impôt local en imposant à leurs administrés une taxe GEMAPI ou prélever une partie de leur budget déjà fort contraint. Rappelons, qui plus est, que cette taxe est assise en partie sur la taxe d'habitation, qui a vocation à disparaître ... Si j'ai bien compris ce que vous avez

L'inquiétude des élus locaux est quelque peu aggravée par la baisse substantielle du budget des agences de l'eau, alors que celles-ci accompagnent les collectivités territoriales dans la prise de compétence GEMAPI et soutiennent leurs actions par le biais de la réalisation d'études et de travaux.

je pense en particulier à la question des digues domaniales, dont la gestion relève principalement de l'intérêt national. Ce transfert placera les intercommunalités dans des situations intenables eu égard au coût considérable qu'elles auront à supporter par rapport aux moyens dont elles disposent, mais aussi aux conséquences parfois tragiques des inondations. Certes, le texte prévoit un rapport sur les effets du transfert de la compétence GEMAPI aux EPCI sur la gestion des fleuves. Mais il eût sans doute été plus constructif et cohérent de légiférer en disposant préalablement des résultats de ce rapport. Aussi ai-je déposé un amendement visant à maintenir d'ores et déjà la responsabilité de l'État en ce qui concerne les digues domaniales, au titre de sa compétence régalienne en matière de sécurité des biens et des personnes. Il semblerait que cet amendement soit irrecevable en application de l'article 40 de la Constitution, car il créerait une charge publique supplémentaire. Je l'entends, mais, à ce stade, si l'échéance du désengagement de l'État en 2024 est confirmée, il y aura bien,

À quelques jours de la nouvelle année et du temps des voeux, permettez-moi, madame la ministre, de souhaiter que le Parlement puisse un jour disposer du temps nécessaire à l'élaboration de lois pertinentes et opérantes, afin d'assurer aux collectivités territoriales la sagesse de la loi, la stabilité des dispositions législatives et la capacité à réaliser les obligations que la loi leur confie. Ces voeux n'empêcheront pas le groupe Union Centriste de voter cette proposition de loi,

à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations, poétiquement appelée compétence GEMAPI. Cette initiative est venue répondre au besoin de gestion intégrée d'une compétence, à la suite de la multiplication des phénomènes d'inondations, notamment dans le Var, à Vaison-la-Romaine, dans l'Aude ou en Bretagne, et de phénomènes extraordinaires, comme la tempête Xynthia, qui ont causé non seulement des pertes humaines, mais également des désastres économiques considérables. Rien que pour les catastrophes survenues dans le Var en 2010 et 2011, on a déploré vingt-sept morts, près de 2 milliards d'euros de dégâts matériels et 35 000 sinistrés, ainsi que 2 000 entreprises et de nombreuses exploitations agricoles touchées. touchées. Lors des débats de la loi MAPTAM, il avait été indiqué que ces catastrophes naturelles provoquaient en moyenne plus de 1 milliard d'euros de dégâts en France. nous savons bien que de tels phénomènes sont malheureusement appelés à se reproduire, avec le réchauffement climatique et la poussée de l'urbanisation, en particulier sur les territoires littoraux où la densité de construction était, en 2010, quatre fois supérieure à la moyenne nationale.

Au regard de ces enjeux majeurs, il paraissait indispensable de définir une compétence ciblée en matière de protection contre les inondations ; une compétence qui permette, d'une part, de clarifier et de coordonner des niveaux de responsabilités jusque-là éclatées- sur 9 000 kilomètres de digues, on dénombre plus de 1 000 gestionnaires différents -et, d'autre part, d'associer deux compétences en une pour une vision plus stratégique des politiques publiques de protection des personnes et des biens, de préservation de la qualité de l'environnement et de maîtrise de l'urbanisation. De fait, avec la loi MAPTAM, l'EPCI à fiscalité propre devient l'acteur incontournable dans la démarche de prévention des risques d'inondation et de submersion, en cohérence avec les actions d'aménagement qu'il mène par ailleurs, comme le PLUI et le SCOT. Pour autant, comme il a déjà été souligné, cette compétence demeure techniquement complexe, et de nombreuses interrogations et inquiétudes émanent des élus locaux. Elles révèlent la difficulté à organiser une structuration institutionnelle adéquate dans les délais réglementaires.

À la veille de l'inscription de la compétence GEMAPI dans les statuts des intercommunalités, la proposition de loi soumise à notre examen offre donc des clarifications et des assouplissements nécessaires, mais pas anodins, sans que les problèmes centraux soient pour autant complètement résolus. soient pour autant complètement résolus. En effet, dans des délais proches de l'urgence, la proposition de loi présente des dispositions qui rassurent les élus locaux et répondent à des problèmes opérationnels.

locaux ; l'extension de l'assistance technique des départements à la prévention du risque d'inondation au titre de la solidarité et de l'aménagement du territoire, ce qui démontre, de manière plus générale, l'importance de la collectivité départementale en la matière l'assouplissement des modalités de transfert ou de délégation de la part des communes ou des EPCI aux syndicats mixtes de droit commun, aux EPTB et aux EPAGE, notamment en termes de sécabilité interne, externe et géographique. Cet assouplissement donnera plus de libertés aux territoires pour définir l'organisation institutionnelle qu'ils jugeront la plus adéquate. Il convient néanmoins de prévenir un émiettement de la compétence, qui nuirait à la cohérence des actions conduites et à l'identification d'un opérateur responsable. Enfin, d'autres mesures, comme la possibilité pour un syndicat mixte ouvert d'adhérer à un autre syndicat mixte ouvert, représentent, selon nous, des avancées. C'est le cas aussi de la clarification du régime des responsabilités, qui demeure néanmoins imparfaite.

Sur ce dernier point, l'introduction de cette nouvelle disposition met en exergue l'incomplétude de la loi, notamment sur le financement de la compétence et l'articulation de celle-ci avec l'ensemble des compétences relevant du cycle de l'eau. relevant du cycle de l'eau. Restent des insuffisances auxquelles il faudra répondre ultérieurement. En effet, au-delà de l'intérêt de cette proposition de loi, et quand bien même elle s'attelle au plus urgent, plusieurs problèmes demeurent,

comme le risque de submersion marine et la lutte contre l'érosion du trait de côte. Je pense aussi à l'articulation avec les compétences « eau et assainissement ». Nous savons en effet que les eaux de ruissellement et l'érosion des sols ont un impact sur les risques d'inondation. la responsabilité des gestionnaires d'ouvrages est encore traitée de manière imparfaite, qui plus est dans un contexte où les missions d'appui technique n'ont manifestement pas mené à terme tous leurs travaux. au financement de la GEMAPI, il ne fait l'objet que d'un rapport du Gouvernement au Parlement, ce qui n'engage pas à grand-chose ... Par ailleurs, le financement en investissement parfois être entravé par la limitation des dépenses de fonctionnement des membres des syndicats mixtes, alors qu'il y va de la sécurité des territoires. nous restons convaincus que le financement proposé n'est pas à la hauteur des enjeux de vulnérabilité des populations évoqués dans mon propos introductif, quand bien même les dispositifs de financement tels que le fonds Barnier perdurent. Une remise à plat du financement du cycle de l'eau s'avère nécessaire pour évoluer vers des logiques de bassin et des solidarités territoriales amont-aval, d'autant plus compte tenu des fortes contraintes financières qui pèsent sur les collectivités territoriales et leurs partenaires, comme les agences de l'eau. À titre indicatif, le Centre européen de prévention du risque d'inondation observe que les travaux réalisés aujourd'hui par les collectivités engagées dans des programmes de travaux, comme les programmes d'action pour la prévention des inondations dans le cadre du plan Submersions rapides, coûtent un peu plus de 1 million d'euros par kilomètre pour ce qui concerne le confortement d'ouvrage, voire 1,7 million d'euros par kilomètre pour l'augmentation du niveau de protection des digues.

Parce que nous souhaitons que la mise en oeuvre de cette compétence se fasse dans des conditions plus sereines et plus durables pour les territoires, nous voterons en faveur de ce texte tout en regrettant, comme d'autres, le délai de réflexion laissé au législateur qui, pour le coup, ne favorise pas- c'est un euphémisme ! -la tranquillité des échanges et ne permet pas d'aborder l'ensemble des problèmes soulevés localement, alors que le risque d'inondation constitue un risque majeur. La

Cette problématique porte en effet de lourds enjeux : des enjeux financiers, comme cela vient d'être rappelé, des enjeux environnementaux, des enjeux en termes de gouvernance et, plus largement, des enjeux de cohérence territoires. La loi MAPTAM de 2014, puis la loi NOTRe de 2015 ont en effet profondément redessiné le périmètre d'action de nos collectivités, sans toujours penser à l'ensemble de leurs conséquences. En proposant d'aménager dans le temps le transfert de la compétence GEMAPI aux EPCI, nos collègues de l'Assemblée nationale ont fait un geste envers nos territoires. Il convient de le souligner et d'en saluer les initiateurs. La date butoir avait déjà été modifiée une première fois, afin de favoriser la continuité de l'exercice des missions Cette nouvelle proposition de loi nous permet d'envisager l'après-2020 pour des territoires qui souhaiteraient continuer à exercer de telles missions. C'est le cas des conseils départementaux. Nombre d'entre eux ont d'ailleurs sollicité leurs parlementaires pour faire connaître leur désir de continuer à s'impliquer dans l'exercice des missions

mon département, la Somme, a été concerné, tant par la submersion marine au début des années 1990 que par les inondations à la fin du siècle dernier, phénomène certainement lié à une crue de nappes perchées, ce qui n'était pas banal et difficile En réaménageant le calendrier de mise en oeuvre de la compétence GEMAPI, cette proposition de loi prête donc l'oreille aux sollicitations des élus de terrain. Dans son article 1, la proposition de loi prévoit la mise en place d'un régime dérogatoire concernant la responsabilité des établissements chargés des structures transférées. Il s'agit d'une mesure de bon sens. Comment imaginer l'inverse ? Il faut que la responsabilité de l'entretien soit progressivement transférée, afin que le rôle de chacun soit clairement identifié. Je crois que cette approche fait l'unanimité. Sur ce point,

Lors des débats en commission, nous avions demandé que les principaux gestionnaires de fleuves, de zones côtières, de digues domaniales et de zones de montagne soient associés à cette concertation. M. le rapporteur et nos collègues de la commission des lois n'ont pas souhaité retenir cette approche. Je crois que le concours de l'ensemble des acteurs du cycle de l'eau est pourtant nécessaire pour résoudre cette problématique fondamentale du financement des missions en matière de GEMAPI. Nous ne pouvons pas faire l'impasse sur ce sujet. Les articles 3 et 4 introduisent un principe de

pour transférer tout ou partie de cette compétence à des établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux, les EPAGE, ou à des établissements publics territoriaux de bassin, les EPTB. La faculté de transférer ces missions consacre de fait le principe de la responsabilité confiée au plus compétent. J'approuve bien entendu les ajustements opérés par la commission des lois.

actions de lutte contre l'érosion des sols. Il s'agit d'une approche large, qui a le mérite de couvrir l'ensemble du sujet, mais il ne faut pas que cet élargissement pertinent affaiblisse les moyens confiés à l'exercice des missions GEMAPI.

Les collectivités territoriales ont déjà été lourdement impactées par ces réformes complexes, dont la compréhension et la concrétisation sur le terrain n'ont pas été chose aisée. Soumises à un rythme effréné de réaménagement de leur fonctionnement et d'absorption des nouvelles compétences, très peu d'intercommunalités ont pu correctement anticiper la prise en charge de la compétence GEMAPI Cette proposition de loi apporte bien des avancées sur lesquelles je reviendrai. Mais était-il raisonnable de se hâter à quelques jours de la date butoir ? Au pire, cela donne une mauvaise loi, au mieux, une loi. C'était d'ailleurs peut-être l'objectif Avant d'évoquer le contenu du texte, je pourrais parler des domaines qu'il escamote. Les questions du trait de côte et de l'érosion marine en sont absentes, ou présentes très marginalement dans une demande de rapport à l'article 2. Il n'est pas non plus question du financement de la compétence GEMAPI.

Les crues de la Seine et de ses affluents en juin 2016 doivent cependant nous interpeller, car nous savons que ces épisodes ont vocation à se reproduire. Nous l'avons bien compris, ce texte vise à procéder aux derniers ajustements de la GEMAPI. Cette question de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est survenue dans le débat public en raison de la violence d'une crue qui a entraîné une prise de conscience. Il faut mettre fin à un modèle où les compétences sont éclatées et les responsabilités sont diluées. S'il était nécessaire que la compétence GEMAPI soit enfin assumée de façon cohérente, le transfert de charges, lui, pour les collectivités locales n'est pas anodin et effraie les élus locaux. L'une des avancées indéniables de la loi MAPTAM fut de donner un cadre et de définir un chef de file- les intercommunalités -, même si nous ne pouvons que regretter le manque de cohérence de ce cadre avec les périmètres hydrographiques des bassins versants, une rivière ne connaissant pas les limites administratives des communautés de communes. La loi NOTRe, quant à elle, a permis de repousser l'échéance au 1janvier 2018. Nous y sommes ! Permettez-moi de vous faire part de mon expérience d'élue locale dont la collectivité a anticipé le transfert de la compétence GEMAPI au 1 janvier 2017. C'est après deux épisodes violents de crues torrentielles en octobre 2012 et juin 2013 que les élus de mon territoire se sont retroussé les manches pour prendre en charge la reconstruction avec des moyens totalement inadaptés, et ce malgré les accompagnements financiers importants Aujourd'hui, demeure un reste à charge important, qui ne peut être absorbé à l'échelle de nos communes et syndicats. La violence de ces événements tragiques nous a tout d'abord poussés à gérer la crise, puis l'immédiate après-crise avec l'urgence de la reconstruction. Nous avons ensuite entamé collectivement une réflexion d'ampleur sur la gestion de notre environnement et les moyens de mieux prévenir ces crues, ainsi que sur la nécessaire mutualisation des moyens et la meilleure façon d'introduire davantage de solidarité entre l'amont et l'aval. a abouti à la transformation de notre PETR en un syndicat de bassin. Ce dernier dispose désormais de capacités d'action nettement renforcées, tant sur le plan financier qu'en termes d'ingénierie. Il fonctionne sur les bases d'une gouvernance partagée.

Je mesure cependant l'inquiétude des élus, qui peuvent avoir le vertige : plus de 9 000 kilomètres linéaires de digues parsèment nos territoires, et ce même si nous savons que la responsabilité de la collectivité gestionnaire est limitée et encadrée. inquiets, parce qu'ils sont occupés à digérer la réforme de l'intercommunalité, qu'ils doivent composer avec des finances contraintes et qu'ils savent le coût des ouvrages concourant à la GEMAPI.

Nous nous retrouvons également dans les précisions bienvenues apportées au régime de responsabilité limitée des gestionnaires d'ouvrages, notamment pour la période transitoire, qui s'ouvrira dans quelques jours. Celles-ci sont de nature à rassurer. Il en va de même de l'exception temporaire de l'interdiction d'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte exerçant une compétence GEMAPI. Nous sommes également attendus sur les modalités de transfert et de délégation de tout ou partie de la compétence GEMAPI, cette fameuse sécabilité interne inscrite à l'article 3.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, cher Mathieu Darnaud, mes chers collègues, corriger les lois NOTRe et MAPTAM sans renoncer à la volonté de réforme, corriger sans bouleverser à nouveau l'organisation des territoires suppose d'entendre les collectivités territoriales et de respecter les principes de notre République décentralisée, ainsi que l'intelligence territoriale. Ces

qui ne saurait constituer un écueil en commission mixte paritaire. Pour aujourd'hui, nous soutiendrons la proposition de loi qui nous est soumise pour redéfinir la répartition de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations et, ainsi, une approche plus globale et nécessaire. Sans doute, ce texte nous oblige-t-il à nous hâter. Mais le rat de La Fontaine ne s'est-il pas lui aussi hâté avec « patience et longueur de temps » pour finalement libérer le lion de ses filets

1janvier prochain et, de manière exclusive, au 1 janvier 2020, question qui pose évidemment des difficultés auxquelles le texte répond. Départements et régions pourront désormais poursuivre leur action en matière de GEMAPI au-delà du 1janvier 2020. C'est parfait ! Ce texte prend mieux en considération les collectivités locales exerçant tout ou partie de la compétence en les laissant évoluer dans un cadre d'action souple à l'heure où celle-ci n'est exercée que par 15 % des EPCI. Nous renouvelons notre confiance aux collectivités : elles disposeront en l'espèce des moyens de contrôler réellement les financements consentis et les modes d'exercice des compétences transférées. les modalités de transfert et de délégation de la compétence à un syndicat mixte sont assouplies avec notamment la « sécabilité » des quatre missions constitutives de cette compétence. Sont ainsi privilégiées des réponses différenciées et opérationnelles aux problèmes rencontrés par nos territoires. Enfin, la commission des lois a maintenu la faculté pour les EPCI à fiscalité propre de transférer tout ou partie des missions à un ou plusieurs syndicats mixtes. Il s'agit chose. Le deuxième point que je souhaite évoquer, c'est la question de la responsabilité de l'EPCI, qui n'a pas été éclipsée. Les communes et EPCI à fiscalité propre compétents deviendront bientôt gestionnaires de digues et autres ouvrages concourant à la prévention des inondations appartenant à d'autres personnes publiques. Ils bénéficieront du régime de responsabilité limitée prévu par le code de l'environnement. Cependant, pour prendre en compte l'incertitude qui subsistait quant à l'application de ce régime dérogatoire au cours de la période transitoire, il a été prévu que la responsabilité dudit gestionnaire ne pourrait être engagée en raison des dommages que l'ouvrage n'aurait pas permis de prévenir, sauf à ce qu'ils soient dus à un défaut d'entretien par le gestionnaire. point, ce texte traite de la question de l'élargissement du périmètre de la compétence GEMAPI à la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, ainsi qu'à la lutte contre l'érosion des sols. Je rejoins sur le fond le rapporteur : de : de nombreuses inondations sont dues au ruissellement plutôt qu'à la crue d'un cours d'eau. Une commune française sur trois est inondable, en partie ou en totalité. En Seine-et-Marne, mon département, ce ne sont pas moins de 4 400 kilomètres de rivières susceptibles de se transformer en rampes de lancement pour d'éventuelles submersions. Devant ce constat et l'ampleur des risques, notre groupe a déposé un amendement d'appel : dans l'attente de la proposition de

pour notre pays, qui manque d'une politique globale de prévention de l'inondation sur l'ensemble du territoire, à l'exception des plans Grands Fleuves, de se contenter d'un assemblage mal coordonné de dispositifs sectoriels, financés trop souvent de manière aléatoire et parfois en concurrence.

entendre. Deux raisons essentielles expliquaient la situation : l'absence d'une gouvernance clairement identifiée de la compétence « prévention de l'inondation » et l'absence de financement pérenne d'une politique de prévention.

loi a ensuite attribué la compétence GEMAPI aux EPCI à fiscalité propre, premier échelon territorial de proximité de taille suffisante pour agir et désormais présents sur l'ensemble du territoire Mais tenant compte du fait que l'échelon pertinent de l'action était le bassin-versant, qui incluait souvent plusieurs EPCI- la loi n'a donc pas non plus oublié cette réalité -, la loi a prévu la possibilité de déléguer à un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau,

« confié à titre exclusif » aux EPCI à fiscalité propre la prévention de l'inondation, laissant entendre par là que tous les anciens acteurs en étaient exclus. Les articles prévoyant que départements et régions et, d'une façon générale,

Vu la complexité du problème, vu la diversité des domaines et des paramètres à prendre en compte, une gouvernance unique et clairement définie est pourtant la première condition de l'efficacité. cela en cause, comme le fait la proposition de loi sous prétexte qu'existent déjà des syndicats, des EPTB, des départements ou des régions en charge d'une partie seulement de la compétence, constituerait une évidente régression. Cela n'a rien à voir avec le respect des libertés locales ou la confiance faite aux collectivités de s'organiser. Voilà l'origine du lobbying mené pour que rien ne change dès la discussion de la loi. chers collègues, je vous en donnerai ! La présente proposition de loi est le dernier épisode de cette offensive. Rien d'étonnant que ce soit « une demande forte exprimée par plusieurs collectivités territoriales », pour reprendre l'exposé des motifs et comme cela a été amplement rappelé ici même. Jusqu'ici, le résultat s'est limité à un report de la mise en oeuvre de la loi de 2016 à 2018. L'échéance échue, sous prétexte d'une insuffisante préparation, on nous propose rien moins que de supprimer l'un de ses apports essentiels : une gouvernance clairement identifiée en charge de la prévention et de protection contre les inondations, dans sa globalité. Est-ce à dire, pour autant, que le texte issu de la loi MAPTAM serait intouchable ? Certainement pas

-et pour le sud du pays. S'y opposer pour d'obscures raisons politico-juridiques, c'est clairement condamner à l'échec toute politique de prévention des inondations dans de nombreuses villes et la moitié du pays.

Pour conclure, je me contenterai de rappeler que, contrairement à ce que pourraient laisser supposer le jour et l'heure d'examen d'un texte aussi lourd de conséquences, la procédure expéditive utilisée,

En attendant mieux, un rapport de l'OCDE estime que la prochaine grande inondation de l'Île-de-France coûtera 40 milliards d'euros. Ces dix dernières années, 50 % des communes françaises ont été affectées par les inondations : il s'agit bien d'un problème général

ses responsabilités » ! La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte de la commission. l'ensemble de la proposition de loi relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Voici quel

Il n'est en effet ni opportun ni juridiquement utile d'étendre cette disposition aux communes dans la mesure où les EPCI à fiscalité propre seront seuls compétents en matière de GEMAPI à compter du 1janvier 2018. Une telle démarche irait à l'encontre du principe irait à l'encontre du principe d'exclusivité de la compétence. J'ai bien entendu que vous souhaitiez vous assurer du fait que les communes isolées qui ne sont pas membres d'un EPCI à fiscalité propre ne soient pas exclues de la possibilité de conventionner avec le département ou la région. Je souhaite vous rassurer sur ce point, puisque le droit en vigueur prévoit explicitement la situation. Le V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales dispose en effet que, « sur le territoire des îles maritimes composées d'une seule commune, les schémas départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans l'obligation de prévoir la couverture intégrale du territoire par des établissements fiscalité propre ». Les communes concernées disposent donc de compétences relevant du bloc communal et pourront conclure des conventions avec le département ou la région sans que la loi ait à le prévoir expressément.

Les syndicats ouverts interdépartementaux et interrégionaux ont démontré toute leur utilité, en portant d'importants investissements d'intérêt général. C'est le cas, dans la région de notre collègue Pascale Bories que je représente ce soir, du Syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer, qui gère, depuis 2003, les ouvrages de protection contre les crues du fleuve et met en oeuvre le plan Rhône.

de poursuivre leur action dans ce domaine, notamment au bénéfice des syndicats mixtes ouverts dont ils sont membres. Tel est l'objet du présent amendement : sans modifier l'esprit de la proposition de loi, il tend simplement à préciser les formes de participation des départements et des régions.

d'instaurer un reversement volontaire par l'EPCI à fiscalité propre ayant perçu la taxe GEMAPI d'une partie de cette taxe, soit au conseil départemental, soit au conseil régional, soit aux deux. La logique d'affectation de la taxe est respectée, car seules les missions GEMAPI pourront être financées par son produit. Toutefois, en autorisant un reversement aux départements et aux régions, la loi reconnaît la logique de solidarité au niveau supra-communautaire et permet à cette solidarité de s'exercer à une échelle adaptée, par exemple celle du bassin-versant. En effet, les recettes fiscales ne sont pas forcément là où les besoins d'investissement sont les plus importants. En conséquence, chaque convention sera amenée à préciser si le financement des missions retenues s'appuie, en tout ou partie, sur la taxe spéciale GEMAPI ou uniquement sur le budget général des collectivités signataires.

des syndicats mixtes auxquels les EPCI auront transféré tout ou partie de leur compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. En effet, de nombreux EPCI ont transféré ou vont transférer tout ou partie des missions GEMAPI à des syndicats mixtes de droit commun ou à des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, ou EPAGE. Lorsqu'un tel transfert de compétence est opéré, il est impératif que le syndicat mixte compétent soit aussi signataire de la convention obligatoire à intervenir entre les parties prenantes, notamment les départements et régions qui poursuivront leur mission GEMAPI au-delà du 1 janvier 2020. Le présent amendement vise donc à régler expressément ce cas de figure, en prévoyant l'intervention obligatoire à la convention du syndicat mixte bénéficiaire d'un transfert de compétence GEMAPI de la part d'un EPCI.

tend à autoriser un EPCI à fiscalité propre à transférer tout ou partie des missions liées à l'exercice de la compétence GEMAPI à un syndicat de communes ou un syndicat mixte. Les syndicats mixtes du secteur de l'eau se sont étonnés d'apprendre qu'ils pourraient être exclus de la convention que le département ou la région aura l'obligation de conclure, en application des dispositions prévues à cet article 1. Cette exclusion leur paraît contestable dès lors qu'ils comptent parmi leurs adhérents des EPCI à fiscalité propre prévoyant déjà de leur transférer l'exercice de certaines missions attachées à la compétence GEMAPI.

La modification proposée dans le texte issu des travaux de la commission des lois du Sénat contribuerait à revenir sur les équilibres, encore récents, établis dans le cadre de la loi NOTRe, ce qui dépasse très largement l'objet de la présente proposition de loi, centrée sur les modalités d'exercice de la compétence GEMAPI. Il s'agit, ici, de traiter de mesures revêtant un caractère transitoire, à savoir la permission octroyée à un EPCI à fiscalité propre, jusqu'au 1 janvier 2020 seulement, de déroger aux dispositions de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, en autorisant l'intercommunalité à déléguer tout ou partie des missions attachées à la compétence GEMAPI à des syndicats mixtes de droit commun. Je vous propose de rétablir le II de l'article 1, tel que voté par l'Assemblée nationale, cette rédaction permettant de conserver les objectifs que nous partageons tous, sur le fond, sans toucher au droit des collectivités locales dans sa portée générale. Il apparaît en effet préférable d'insérer les dispositions concernées au sein de l'article 59 de la loi MAPTAM, qui traite d'autres mesures transitoires, plutôt que de les inscrire dans le code général des collectivités le III de cet article 1, qui prévoit la possibilité pour les EPCI à fiscalité propre de délibérer pour transférer tout ou partie de la compétence GEMAPI à un syndicat mixte avant la date effective du transfert de compétence, soit avant le 1 janvier 2018. En 2015, le législateur avait pris soin de supprimer la disposition permettant aux régions de contribuer au financement des opérations d'intérêt régional des départements, des communes ou de leurs groupements. Réintroduire des dispositions conférant une faculté de financement encore plus large serait contraire aux objectifs de rationalisation et de diminution des financements croisés. Il n'est donc pas souhaitable, dans un souci de clarification de la répartition des compétences entre les différents échelons des collectivités locales, d'étendre aux régions les dispositions de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, qui est un article de portée générale, et ce même si la disposition envisagée concerne la seule compétence GEMAPI. Il convient également de rappeler que les dispositions introduites à l'article 1 de la présente proposition de loi permettent d'ores et déjà à l'ensemble des régions de poursuivre leur intervention en matière de GEMAPI, ce qui justifie d'autant moins le recours à une modification de cet article L. 1111-10.

La nouvelle rédaction paraît trop restrictive sur la question du financement de la GEMAPI par les régions. Ces dernières pourraient la financer uniquement pour les maîtrises d'ouvrage assurées par une commune, un EPCI ou un syndicat mixte fermé. Or, actuellement, la région Grand Est, tout comme d'autres régions de France- PACA, notamment -, finance ses dispositifs « Eaux et milieux aquatiques » de nombreuses structures, notamment des associations et des syndicats mixtes dits « ouverts ». Par cet amendement, il est donc proposé une formulation plus large, afin que les modalités actuelles de financement de cette compétence

a adopté un amendement tendant à permettre à la région de verser des contributions financières aux projets mis en oeuvre pour l'exercice de la compétence GEMAPI et sous la maîtrise d'ouvrage d'une commune, d'un EPCI à fiscalité propre ou d'un syndicat mixte. Le présent amendement a pour objet d'étendre cette possibilité aux départements, ce qui semble cohérent compte tenu de l'implication de ce niveau de collectivité territoriale dans l'exercice de la compétence GEMAPI, pouvant revêtir différentes formes : la possibilité, prévue à l'article 1, de continuer à exercer directement certaines missions relevant de cette compétence, une assistance technique aux collectivités concernées ou encore une contribution financière à la réalisation de certains projets. S'agissant de cette dernière possibilité, il me semble opportun de mentionner clairement que les projets relevant de la compétence GEMAPI sont susceptibles de recevoir des aides du département, la rédaction de l'alinéa 1 de l'article L. 1111-10 du code général des

pourrait considérer comme illégale une subvention versée par le département à un syndicat mixte compétent pour exercer certaines missions relevant de la compétence GEMAPI.

Les syndicats mixtes ouverts seront exclus de fait du dispositif et ne pourront donc pas bénéficier de ces aides, alors que de nombreux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau ou d'établissements publics territoriaux de bassin auront précisément Comment justifier une telle exclusion ? En l'absence de modifications, la région ne pourra pas financer un syndicat mixte ouvert comptant, notamment, un département parmi ses membres.

par la loi à conclure une convention dont, selon cette même loi, seul un EPCI peut être partie prenante, aux côtés des départements et des régions. Pour nous en tenir à la seule compétence GEMAPI, je rappelle que les articles L. 566-12-1 et L. 566-12-2

EPCI compétents en la matière. Il en va de même des paragraphes II, III et IV de l'article 59 de la loi MAPTAM, dans lesquels viendraient s'insérer les dispositions prévues à l'article 1 Enfin, la commission des lois ne veut pas insulter l'avenir. Il n'est pas impossible que d'autres communes soient à l'avenir dispensées d'adhérer à un EPCI, des communes nouvelles que le législateur jugerait aptes à assumer elles-mêmes les compétences normalement dévolues à l'intercommunalité des communes de la métropole du Grand Paris,

d'une participation à un syndicat mixte ouvert ou à un autre groupement peuvent poursuivre leur action au-delà de 2020. Il me semble- mais je m'interroge encore sur ce point -que cet amendement est entièrement satisfait par l'article 1.

rectifié vise à prévoir qu'un syndicat mixte auquel a été transféré l'exercice de la compétence GEMAPI est partie à la convention conclue entre le département ou la région et l'EPCI compétent. Cette proposition nous semble superflue, puisque les départements et les régions pourront de fait adhérer à de tels syndicats mixtes. En outre, il est préférable que cette convention, qui touche à la répartition des compétences entre les différents niveaux de collectivités, soit conclue avec le titulaire de la compétence GEMAPI, à savoir la commune ou l'EPCI, même si l'exercice de cette compétence a été transféré ou délégué à un syndicat. Ce sera donc une demande de retrait ou, à défaut, un avis

tout ou partie de la compétence GEMAPI à un syndicat mixte. Il entretient une certaine confusion avec les dispositions de l'article 4, qui offrirait cette possibilité de manière permanente en cas de délégation à un EPAGE ou un à EPTB.

y compris par une délibération prise avant le 1 janvier 2018. Cela n'aurait pas grand sens, étant donné que la présente proposition de loi n'entrera en vigueur, au mieux, que dans les derniers jours de 2017. Je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler l'article 2 du code civil : « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. » La commission des lois a observé que les délibérations prises par les EPCI, antérieurement au transfert vers ces structures de la compétence GEMAPI, aux fins de transférer ou déléguer cette compétence avaient peu de chance d'être annulées, compte tenu de la jurisprudence conciliante du Conseil d'État au sujet des actes Néanmoins, puisque la volonté du Gouvernement et de l'Assemblée nationale est d'écarter tout risque d'annulation, la seule solution disponible est de valider expressément par la loi ces délibérations,

Tout comme certains amendements précédents, ils nous apparaissent superflus puisqu'une région peut tout à fait adhérer à un tel syndicat, auquel cas elle devra lui verser une contribution financière annuelle. Ce sera donc une

constitué uniquement d'EPCI et, éventuellement, de communes doit être considéré comme un groupement de communes au sens de cet article. Quant au syndicat mixte ouvert, les départements, comme nous venons de le signaler pour les régions, peuvent tout à fait y adhérer. Ce sera donc une demande de retrait ou, à défaut, un avis défavorable.

vous proposez, en une seule et même disposition, de supprimer la possibilité donnée aux départements et aux régions d'agir dans le domaine de la GEMAPI au-delà du 1 janvier 2020, de supprimer la possibilité donnée aux régions de contribuer au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements et, enfin, de supprimer le régime de responsabilité aménagée pour les EPCI dans le cas de la gestion des digues et des autres ouvrages de protection. Le Gouvernement ne peut vous rejoindre que sur votre souhait de ne pas étendre aux régions les dispositions issues de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales. Il a d'ailleurs déposé un amendement en ce sens. Il ne peut en revanche suivre la proposition de suppression des souplesses que les députés ont adoptées, avec l'accord du Gouvernement, pour faciliter l'exercice de la compétence GEMAPI. Il en est ainsi de la possibilité donnée aux départements et aux régions d'agir dans le domaine de la GEMAPI au-delà du 1 janvier 2020. Certaines de ces collectivités, parfois engagées de longue date dans la prévention des inondations, pourraient ainsi venir en soutien aux actions des intercommunalités. Il en va de même de la disposition relative à la responsabilité des EPCI. Vous proposez de la supprimer, alors qu'il nous paraît au contraire essentiel à la réussite de ce transfert de compétences d'encadrer du mieux possible la responsabilité des acteurs locaux, dans un souci de sécurité juridique. C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur votre amendement. Le Gouvernement

dans le cadre de la convention prévue à l'article 1 de la proposition de loi, à reverser une partie du produit de la taxe GEMAPI au profit des départements et des régions. Le Gouvernement n'est pas favorable à cette mesure. La poursuite volontaire de l'intervention, d'ores et déjà en cours, des départements et des régions au titre de la GEMAPI est permise, permise, mais cela ne remet pas en cause le fait que l'échelon intercommunal devienne, à partir du 1 janvier 2018, le seul titulaire de la compétence à titre obligatoire. Ainsi les EPCI à fiscalité propre doivent être les seuls habilités à instituer une taxe destinée à financer une de leurs compétences obligatoires et à déterminer l'usage qu'ils souhaitent en faire, par exemple pour financer des ouvrages.

aux régions les dispositions de l'article L.1111-10 du code général des collectivités territoriales, qui réserve à ce jour aux seuls départements la faculté de contribuer au financement de projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements.

Le Gouvernement a le souci de maintenir la clarification de la répartition des compétences entre les différents niveaux de collectivités territoriales voulue par le Parlement

permettant aux régions de financer des opérations conduites par les départements, les communes et leurs groupements. Réintroduire aujourd'hui des dispositions conférant une faculté de financement encore plus large serait contraire aux objectifs de rationalisation.

afin de prévoir explicitement que les départements puissent contribuer au financement des projets mis en oeuvre dans le cadre de l'exercice de la compétence GEMAPI, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une commune, un EPCI

jour, monsieur Collombat. Je voudrais lever toute ambiguïté : il n'est pas question d'interdire aux départements et aux régions d'apporter leur contribution à la lutte contre l'inondation. Le problème porte sur les modalités.

l'eau, il est nécessaire de s'assurer que toutes les missions du grand cycle de l'eau sont mises en oeuvre pour atteindre les objectifs notamment de la directive-cadre sur l'eau, de la directive inondation et de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin, et une gestion intégrée de l'eau au coeur de l'aménagement et du développement durable des territoires. programmer et à planifier, dans un délai de cinq ans, l'exercice de ces nouvelles missions, pour assurer une vision à moyen terme et une cohérence globale

notamment les EPCI à fiscalité propre, auront déjà fort à faire au cours des prochaines années pour assumer leurs nouvelles compétences en matière de GEMAPI. L'adoption de cet amendement risquerait de créer une lourdeur supplémentaire. En outre, En outre, plusieurs autres missions mentionnées à l'article L. 211-7 du code de l'environnement feront nécessairement l'objet d'une réflexion dans le cadre de la GEMAPI l'exploitation des ouvrages hydrauliques existants, la maîtrise des eaux de ruissellement, la lutte contre la pollution des eaux. L'amendement semble donc de faible portée. Enfin, cette proposition de loi a pour objet de faciliter l'exercice de la compétence GEMAPI et non de traiter de l'ensemble de la politique de l'eau.

prévoit la mise à disposition de l'EPCI compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, des ouvrages ou infrastructures qui appartiennent à une personne morale de droit public, ouvrages qui n'ont pas pour vocation exclusive la prévention des inondations ou des submersions, mais sont de nature à contribuer à cette prévention, eu égard à leur localisation et à leurs caractéristiques. Cet amendement se veut donc protecteur des intérêts des EPCI sur lesquels pèseront toutes les responsabilités en matière de protection des populations les systèmes d'endiguement. Certes, un régime de responsabilité limitée a été introduit par la présente proposition de loi durant la période transitoire. Mais ce mécanisme de responsabilité limitée, même s'il constitue une avancée appréciable, reste néanmoins insuffisant selon les spécialistes. En effet, l'EPCI peut se voir mettre à disposition un ouvrage de nature à contribuer à la prévention des inondations, qui n'aura pas fait l'objet d'un entretien suffisant ou de travaux de remise en état au préalable. Or, à défaut de contraindre le propriétaire à exécuter les travaux nécessaires ou à prévoir une participation de sa part, la charge complète de la mise aux normes de ces ouvrages pèsera sur le seul EPCI.

Nous avons rejeté cet amendement en commission. Rappelons que le principe selon lequel les ouvrages concourant à la prévention des inondations sont mis à la disposition des communes ou des EPCI compétents n'a pas pour effet, en lui-même, de faire peser sur les communes ou EPCI le poids de la remise en état des ouvrages lorsque ceux-ci ont été mal entretenus ou lorsqu'ils ne sont plus plus conformes à la réglementation. La commune, ou plus généralement l'EPCI, sera maître de décider quels ouvrages il entend faire autoriser par l'État. Les ouvrages autorisés devront être entretenus et, éventuellement, réaménagés conformément aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation par leur gestionnaire, c'est-à-dire par l'EPCI- ou, en pratique, par un syndicat mixte auquel il aura transféré ou délégué cette charge. Les dépenses d'aménagement, d'entretien et de surveillance incomberont donc à l'EPCI. En revanche, les ouvrages non autorisés ne seront plus considérés comme des digues ou des ouvrages concourant à la prévention des inondations. L'EPCI n'en sera donc plus gestionnaire. Il appartiendra à leur propriétaire de les « neutraliser », c'est-à-dire de les araser ou d'y percer une brèche, pour qu'ils n'entravent pas l'écoulement des eaux.

En effet, cet amendement vise des ouvrages qui ne sont pas des digues et dont l'état d'entretien correspond à l'usage qui en est normalement fait, et pas spécifiquement à un objectif de prévention des inondations. Le principe, instauré par la loi MAPTAM au moment de la création de GEMAPI, des mises à disposition au profit des EPCI exerçant leur compétence, des infrastructures pouvant contribuer à la mission de prévention des inondations- par exemple un remblai ferroviaire -est celui de l'absence de coût pour le propriétaire de l'infrastructure, par exemple la SNCF. La logique de ce principe est qu'il n'incombe pas aux propriétaires d'infrastructures d'exercer les missions de protection contre les inondations. Par ailleurs, s'agissant du supposé mauvais état des infrastructures qui seraient mises à disposition, il convient de rappeler deux points essentiels. En premier lieu, le bon état à atteindre pour assurer la fonction d'infrastructure n'est pas forcément le même que pour assurer une fonction très spécifique de protection contre les inondations. En second lieu, l'EPCI à fiscalité propre reste libre de déterminer le niveau de la protection qu'il entend offrir aux territoires. Ainsi, dans le cas où un ouvrage serait repris en gestion dans un état initial qui ne satisferait pas l'EPCI, celui-ci pourrait néanmoins l'inclure dans un système d'endiguement après en avoir expertisé les caractéristiques. Dans ce cas, le niveau de protection sur lequel l'EPCI

L'EPCI pourra par la suite engager librement et à son rythme les travaux d'amélioration aux fins d'offrir à la population un niveau de protection supérieur. Il convient par ailleurs Il convient par ailleurs de rappeler que ces travaux d'amélioration, s'ils sont effectués dans le cadre d'un plan d'action de protection des inondations, peuvent bénéficier d'un financement de la part du fonds Barnier,

En effet, son objet est de permettre à un EPCI qui perçoit la taxe GEMAPI d'utiliser une partie du produit de cette taxe pour financer des investissements à réaliser sous maîtrise d'ouvrage départementale ou régionale en matière de GEMAPI. L'intérêt de cet amendement est de sécuriser l'utilisation qui peut être faite du produit de cette taxe par les EPCI. En effet, sans la base légale proposée par cet amendement, les EPCI ne pourront pas, sans risque contentieux, financer par des subventions des actions GEMAPI menées sous maîtrise d'ouvrage départementale ou régionale. En résumé, il s'agit de sécuriser des accords financiers que les conventions vont inévitablement prévoir si elles coopèrent à l'échelle d'un bassin-versant, voire tout au long d'une rivière principale. dans ce domaine, les oppositions aux travaux prévus sont nombreuses. Et quand les opposants à un projet sont à court d'arguments techniques, ils cherchent inévitablement des arguments juridiques et financiers.

L'article 1de la présente proposition de loi permet aux départements et aux régions assurant une ou plusieurs des missions attachées à la compétence GEMAPI de poursuivre leurs engagements en la matière au-delà du 1janvier 2020. Cet amendement vise, à l'heure où certains départements connaissent des difficultés à affecter leur part de taxe d'aménagement, à permettre expressément à ceux qui le souhaiteraient, sans faire naître d'obligation en la matière ni de charge supplémentaire, d'utiliser une partie de celle-ci pour financer des dépenses en matière de GEMAPI. À l'heure actuelle, certaines dépenses en matière de milieux aquatiques peuvent déjà être financées par la taxe d'aménagement. Il n'en va pas de même pour les dépenses relatives à la protection contre les inondations ou les coulées d'eaux boueuses après orage. Or ce sont les opérations les plus coûteuses et les plus nécessaires à la protection des populations qui émargent sur cette mission.

Cet amendement prévoit d'inclure les dépenses liées à l'exercice de missions relevant de la GEMAPI parmi celles auxquelles peut être affecté le produit de la taxe d'aménagement perçue par les départements. Néanmoins, cette proposition de loi n'a pas pour objet d'étendre le domaine d'intervention des départements et des régions dans le domaine de la GEMAPI, mais de permettre à ceux qui le souhaitent de continuer à oeuvrer

: La parole est à M. Jérôme Bignon. Si la compétence GEMAPI permet d'assurer la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations sur tout le territoire national, elle ne permet pas d'assurer, aussi bizarre que cela puisse paraître, la cohérence des actions à l'échelle adaptée du bassin-versant de manière homogène- et Dieu sait si celui-ci est essentiel en matière d'écoulement des eaux -ni d'assurer l'exercice de certaines missions en subsidiarité à l'échelle adaptée hydrographique. Cet amendement vise donc à demander aux collectivités territoriales d'identifier les actions d'intérêt commun à l'échelle hydrographique qui nécessitent une implication à une échelle supra-administrative, souvent interdépartementale ou interrégionale, qui seront portées dans le cadre d'un ou de plusieurs projets d'aménagement d'intérêt commun, mis en oeuvre par un établissement

est à M. Stéphane Artano, sur l'article. Je souhaite attirer l'attention de la Haute Assemblée sur les conséquences du transfert de la GEMAPI au bloc communal, dans les territoires ultramarins, et plus particulièrement à Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans l'archipel, il n'y a que deux communes, et l'intercommunalité ne trouve pas à s'appliquer quand il s'agit de mettre en commun des moyens entre deux îles. Au-delà des modifications qui font l'objet de cette proposition de loi, je formule une question simple : qui assurera l'exercice de la compétence GEMAPI, obligatoire à Saint-Pierre-et-Miquelon Ce territoire est exposé aux aléas météo-marins et subit à la fois les impacts des dépressions subarctiques et des cyclones remontant la côte nord-américaine. Si je mets de côté la gestion des milieux aquatiques terrestres, les territoires ultramarins tels que Saint-Pierre-et-Miquelon ne pourront pas faire face aux coûts insurmontables de protection et d'entretien de leur littoral. Ils ne disposent en effet pas de moyens suffisants, qu'ils soient financiers, humains ou matériels. Ces petites communes ne peuvent gérer seules les enjeux du réchauffement climatique. C'est pourquoi l'État doit continuer à exercer une compétence générale en la matière. était le sens de deux amendements que j'avais déposés, mais qui ont été jugés irrecevables au titre de l'article 40 de la constitution. La question qu'ils soulèvent est pourtant cruciale. Prenons l'exemple de l'île de Miquelon-Langlade, qui compte 500 habitants. Aujourd'hui, par laxisme, l'État n'intervient pas et laisse les assauts de la mer entrer au sud du village et menacer des habitations. Demain, la mairie devra-t-elle assumer ce désengagement préjudiciable de l'État ? C'est inacceptable. De plus, l'article 1530 du code général des impôts relatif à la taxe GEMAPI ne sera pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, car c'est la collectivité territoriale qui est compétente en matière Preuve que cette question est complexe : Mme le maire de Miquelon-Langlade a écrit, mi-septembre, au Gouvernement sur la base des arguments que je viens de développer. elle n'a pu avoir les éclaircissements nécessaires que son courrier appelait. Je me fais donc son relais, dans cet hémicycle : Mme la ministre, pouvez-vous apporter des éléments de réponse à ces élus et, à travers eux, aux habitants de Saint-Pierre-et Miquelon ?

? La précision proposée dans le présent amendement est intéressante, bien que je me demande à quoi renvoie exactement la notion de « territoires ruraux non urbanisés La deuxième phrase de l'article 2 précise que ce rapport présente « un bilan de la protection du territoire national contre les risques d'inondations fluviales et de submersion marine et étudie notamment les évolutions institutionnelles et financières

la question suivante : quel est l'échelon le plus pertinent pour exercer la compétence GEMAPI dans les outre-mer ? De plus, si l'article 40 de la Constitution a été opposé aux autres amendements que nous avons déposés, qu'en est-il de l'article 72-2 de la Constitution, en vertu duquel « tout transfert de compétence entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice »

messieurs les sénateurs, je vous propose de revenir sur la rédaction de l'article 3 du présent texte. En effet, il n'est pas souhaitable de déplacer dans le code général des collectivités territoriales des dispositions visant spécifiquement les modalités d'exercice de la compétence GEMAPI par des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, les EPAGE, ou des établissements publics territoriaux de bassin, les EPTB. Ces deux types de structures spécifiques, constituées sous forme de syndicats mixtes ouverts, font l'objet d'une définition précise précise à l'article L. 213-12 du code de l'environnement. Il convient de maintenir rassemblées au sein de ce même article l'ensemble des dispositions s'y rapportant spécifiquement. En effet, dans sa version actuelle, le présent article aboutirait à proposer deux rédactions différentes

pour les acteurs appelés à les mettre en application. En résulterait, potentiellement, une insécurité juridique. La rédaction proposée à travers le présent amendement permet d'éviter cet écueil. Par ailleurs, il convient de supprimer la référence faite aux missions mentionnées au I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, dans la mesure où cette mention aurait pour effet d'élargir le principe d'une sécabilité interne à l'ensemble des missions relatives à la gestion de l'eau. Une telle

rencontrées sur le terrain. Par son I, le présent amendement tend à remédier aux problèmes susceptibles d'être soulevés par la suppression des termes « de gestion de l'eau et des cours d'eau » à l'alinéa précédent.

Quant aux dispositions des alinéas 5 à 9, elles ont le même but que les II et III de l'article 1 du texte de la proposition de loi issu de la première lecture à l'Assemblée nationale,

et, d'autre part, celle de délibérer pour transférer tout ou partie de cette compétence à des syndicats mixtes de droit commun, avant d'en être titulaires, avant le 1 janvier 2018. Compte tenu de

Enfin, le Gouvernement souscrit à la nécessité de permettre une sécabilité géographique par délégation aux EPAGE et EPTB. Je relève que cette sécabilité géographique est déjà autorisée par transfert

Gouvernement, il serait inopportun d'insérer dans le CGCT les dispositions relatives au transfert et à la délégation de la compétence GEMAPI à un EPAGE ou un EPTB, au motif que ces dispositions dérogent au droit commun. Toutefois, le Gouvernement nous propose de maintenir dans le CGCT des dispositions tout aussi dérogatoires, ce qui concerne le transfert de la compétence GEMAPI à un syndicat mixte de droit commun, avec une sécabilité géographique et fonctionnelle. Au contraire, et par cohérence, la commission a jugé préférable de regrouper au sein d'un même code toutes les règles relatives au transfert et à la délégation de la compétence GEMAPI, quel

le Gouvernement nous reproche d'avoir étendu à l'ensemble des missions relevant de la politique de l'eau les possibilités de transfert partiel de compétences, au lieu de les circonscrire à la seule GEMAPI. Mais le texte de l'Assemblée nationale opérait un recul par rapport au droit existant en vigueur, dans le domaine de la gestion de l'eau, un EPCI peut d'ores et déjà transférer ses compétences à un syndicat sur une partie seulement de son territoire, ou à plusieurs syndicats sur des parties distinctes de son territoire. commission va un peu au-delà du droit en vigueur : elle ouvre la voie, en cas de transfert, à la sécabilité interne de toutes les missions relevant de la politique de l'eau. Je vois mal pourquoi cette sécabilité interne serait bienvenue en matière de GEMAPI et malvenue dans les autres domaines de la politique de l'eau, d'autant que les différentes missions énumérées

Mais je dois vous avouer que le présent amendement nous a laissés perplexes. La notion de délégation, employée dans cette proposition de loi, est parfaitement claire. Elle répond à la définition figurant à l'article L. 1 111-8 du code général des collectivités territoriales, à cette seule différence que, en matière de GEMAPI,

une certaine confusion. Cet amendement est présenté comme rédactionnel, alors qu'il vise à modifier le fond du droit. À l'instar de l'Assemblée nationale, la commission a souhaité que la délégation de tout ou partie de la compétence GEMAPI à un syndicat mixte de droit commun, c'est-à-dire un EPAGE ou un EPTB, ne soit possible que pour une période courant jusqu'au 1 janvier 2020. Or, avec cet amendement, les délégations votées avant 2020 continueraient d'être valables passé cette date. Enfin, contrairement à ce qui est indiqué dans l'objet de cet amendement, il ne s'agit pas de la possibilité, pour un syndicat mixte, d'adhérer à un autre syndicat mixte

la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, la lutte contre l'érosion et l'extension éventuelle de la compétence GEMAPI à ces sujets.

Pour autant, c'est le lien entre la gestion des eaux pluviales et l'assainissement que le Gouvernement entend maintenir. À nos yeux, il n'est pas souhaitable d'étendre le champ de la compétence GEMAPI au-delà des quatre items mentionnés au I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. Les missions liées à la maîtrise des eaux pluviales et du ruissellement doivent donc, selon le Gouvernement, rester partagées entre les différents échelons de collectivités territoriales. En effet, et conformément à la jurisprudence du Conseil d'État,

et potentiellement à la taxe GEMAPI, les investissements liés à un éventuel sous-dimensionnement des équipements de gestion des eaux pluviales. En revanche, les équipements structurants permettant de faire face aux risques d'inondations consécutives de pluies d'intensité exceptionnelle relèvent bien de la compétence GEMAPI, au titre des items 1 et 5 de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. Ces équipements peuvent donc être financés par le produit de la taxe GEMAPI.

des départements ont une expertise complémentaire à faire valoir dans le domaine : il est utile qu'ils puissent la mettre à disposition des communes et des EPCI qui la solliciteraient. Laissons aux élus municipaux et intercommunaux le choix entre les prestations

d'acteurs incontournables des politiques de l'eau dans les marais. Sans eux, notre économie, nos paysages et notre environnement seraient profondément altérés.

apparaît donc contestable. En effet, en instituant la compétence GEMAPI, le législateur n'a pas voulu exonérer les propriétaires riverains de cours d'eau non domaniaux de leurs obligations d'entretien des cours d'eau- curage, enlèvement des embâcles et débris, etc. Ces obligations sont la contrepartie de leur droit de propriété sur le lit du cours d'eau, qui emporte le droit d'en extraire des matériaux ; d'un droit d'usage préférentiel de

Gouvernement est identique. Je veux vous expliquer que le paiement de la redevance est directement lié au statut de propriétaire des membres de l'ASA, qui paient pour le fonctionnement de leur association. Il n'y a donc pas d'inégalité devant l'impôt dans la mesure où ces contribuables ne sont pas dans la même situation. En l'espèce, il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait de payer cette redevance et le fait d'être assujetti à la taxe GEMAPI. En outre, votre amendement prévoit un crédit d'impôt sur le revenu et donc grève le budget de l'État : une telle mesure relève en principe de la loi de finances. Toutefois, il est possible qu'existent localement des regroupements entre les missions dévolues aux intercommunalités du fait de la compétence GEMAPI et celle qui est assurée par les ASA.

Le premier motif tient aux finances publiques. La taxe GEMAPI, prévue à l'article 1530 du code général des impôts, taxe affectée, est destinée à permettre aux EPCI à fiscalité propre, qui seront les seuls à compter du 1 janvier 2018 à devoir exercer de manière obligatoire la compétence GEMAPI, de bénéficier de moyens de financement suffisants. Aussi, dans la mesure où il s'agit d'une taxe affectée au financement exclusif de la compétence GEMAPI, toute extension de son champ de financement ne saurait être opérée sans une extension du champ de compétence GEMAPI défini dans le code de l'environnement. On vient il est impossible de prévoir cette extension, sans remettre en cause le caractère affecté de cette taxe. Le second motif est lié à la compétence GEMAPI elle-même.

pour financer une compétence telle que la maîtrise des eaux pluviales ou du ruissellement, qui demeure partagée entre toutes les collectivités territoriales, au titre du code de l'environnement. J'attire en outre votre attention sur un point important la gestion de fortes pluies est déjà couverte, comme je l'ai indiqué précédemment, par le 1° et le 5° de la compétence GEMAPI lorsque celles-ci sont susceptibles d'engendrer des inondations. inondations. Ainsi, dans les cas de bassins versants agricoles présentant des enjeux de ravinement, d'érosion et de pollution, qui jouent un rôle majeur dans les phénomènes de ruissellement, certaines infrastructures de stockage en amont peuvent d'ores et déjà être financées par la taxe GEMAPI, au titre de la prévention des inondations. du code de l'environnement était rattaché à la compétence GEMAPI et non plus à la compétence assainissement, conformément à la jurisprudence de la Communauté européenne, cela poserait la question de la gestion des installations qui traitent à la fois les eaux usées et les eaux pluviales, comme les réseaux unitaires de transport des eaux ou certains bassins d'orage ayant une vocation à la fois de récupération des eaux de pluie et de stockage des eaux usées en prévention des débordements du réseau et de la station d'épuration, qui relèvent logiquement de la responsabilité de la collectivité compétente au titre de l'assainissement. De plus, la problématique de la gestion des rejets d'eaux pluviales dans les milieux aquatiques ne serait plus abordée sous l'angle qualitatif si le 4° de si le 4° de l'article précité était rattaché à la compétence GEMAPI. Or cet aspect doit être assuré, conformément aux exigences de la directive-cadre sur l'eau. L'ensemble de ces éléments me conduisent à constater l'inopportunité de l'article 9, que je vous demande de bien vouloir supprimer. Ce sera

taxe, dans des proportions limitées d'ailleurs, ne revient pas à remettre en cause sa nature de taxe affectée. Ensuite, personne n'est exposé au risque de double paiement. La commission n'a pas relevé le plafond de la taxe ; elle a seulement permis aux communes et EPCI d'en faire le meilleur usage pour prévenir les inondations et gérer les milieux aquatiques. Enfin, l'article 9 serait contraire à la politique défendue par le Gouvernement en matière d'incitation à la mise en place de solutions de rétention des eaux à la source par la désimperméabilisation ou la végétalisation des surfaces. Mais la commission n'a nullement prévu que la taxe GEMAPI doive être intégralement affectée à la construction de canalisations. Tout au contraire, nous avons rappelé dans le rapport que la prévention des inondations liée au ruissellement passait aujourd'hui non plus par le « tout-tuyau », mais par différents types d'action et de travaux, tels que le terrassement, le creusement de noues et de fossés, le changement de revêtement de la voirie, la plantation de haies, la végétalisation, l'urbanisation raisonnée. En revanche, je suis heureux d'entendre Mme la ministre affirmer que certains équipements de maîtrise du ruissellement peuvent déjà être financés par la taxe GEMAPI, au titre des missions d'aménagement d'un bassin hydrographique et de prévention des inondations. D'après ce que nous avons entendu dire lors des lors des auditions, les préfets sont loin d'être tous du même avis. On leur écrira ! Les élus locaux pourront désormais se prévaloir des propos tenus ici même par vous, madame la ministre, en séance publique, qui plus est. Il serait d'ailleurs utile que vous précisiez quels types de travaux sont d'ores et déjà éligibles, sans qu'il soit

Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des raisons qui me conduisent à être en désaccord avec ce texte, qui met à mal l'un des aspects fondamentaux de la loi dite GEMAPI.

! Par ailleurs, n'est pas non plus prise en compte la vision géophysique de l'eau, dont les frontières ne sont pas administratives. Le concept de bassins versants est plus large que le simple concept de bassins versants agricoles évoqué par Mme la ministre. La géographie de l'environnement ne fait pas encore bon ménage, me semble-t-il, avec le droit des collectivités territoriales.

de la mise en oeuvre du transfert de compétence, je confirme que cette proposition de loi est utile : elle rassure et elle simplifie. Aussi, le groupe Union Centriste votera à l'unanimité cette proposition de loi.

Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité (procédure accélérée)